Madame la présidente, monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, mardi dernier, deux surveillants ont été grièvement blessés par un détenu et sa compagne dans une unité de vie familiale de la maison centrale de Condé-sur-Sarthe. Nos pensées vont d'abord vers ces hommes et vers leurs familles. Ils ont vécu dans leur chair cette attaque que vous avez vous-même qualifiée, madame la garde des sceaux, de terroriste. Et il s'agit bien de cela Au-delà, comme en témoignent les mouvements devant certains établissements hier et ce matin, l'émotion est vive parmi les personnels pénitentiaires. Elle est bien sûr légitime. À ces femmes et à ces hommes qui, derrière les murs de nos prisons, exercent au quotidien un métier difficile, méconnu de nos concitoyens et pourtant essentiel à la sécurité de notre pays, je veux exprimer la gratitude et le respect de la représentation nationale. Depuis dix-huit mois, le Gouvernement a beaucoup agi pour les personnels pénitentiaires. Cette ambition se manifeste notamment dans le projet de loi de programmation 2019-2022 et de réforme pour la justice défendu devant le Parlement depuis l'automne, qui prévoit à la fois des moyens pour l'administration pénitentiaire sur les quatre années à venir, une réforme du sens et de l'efficacité des peines, et des mesures qui doivent permettre de renforcer la sécurité des personnels de surveillance et des établissements. Madame la garde des sceaux, au-delà de cet effort budgétaire, qui est nécessaire, et de ces mesures, pouvez-vous nous dire ce qui a déjà été entrepris et surtout ce que vous comptez faire pour améliorer encore la sécurité de nos prisons

lors de l'attaque terroriste qui a eu lieu à Condé-sur-Sarthe. Je tiens à témoigner devant vous de leur professionnalisme et de leur courage face à une attaque d'une rare violence ; nous devons leur rendre hommage, ainsi qu'aux forces de sécurité qui ont mis fin à cette attaque. Une enquête judiciaire est en cours et, de mon côté, j'ai saisi l'Inspection générale de la justice pour analyser les conditions dans lesquelles cette attaque a pu intervenir.

nous posant un certain nombre de questions. Les procédures de fouille des visiteurs, en particulier dans ces établissements sécuritaires, sont-elles adaptées ? Les moyens techniques permettant de détecter les objets métalliques peuvent-ils être améliorés et renforcés ? des détenus sont-ils bien pris en compte pour assurer leur affectation, notamment dans le cadre de l'accès aux unités de vie familiale ? Depuis dix-huit mois, vous l'avez rappelé, monsieur le sénateur, notre gouvernement a agi pour renforcer la protection des personnels de surveillance. Nous avons en effet décidé de recruter 1 100 personnes supplémentaires chargées de la surveillance. Nous avons renforcé les effectifs du renseignement pénitentiaire. Nous avons amélioré les équipements de sécurité des surveillants pénitentiaires.

en lien avec les organisations syndicales, que je recevrai très prochainement à ce sujet. Bien sûr, j'entends les impatiences et je les comprends, mais soyez certains que la résolution du Gouvernement est absolument sans faille. faille. La sécurité de nos établissements et de nos personnels est une condition qui n'est pas négociable et nous y travaillons activement. Social Européen. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation. Mardi dernier, le quotidien titrait : « Aides européennes pour le secteur rural : la France va-t-elle perdre ses millions ? » Cette interrogation fait suite au constat de sous-consommation du fonds qui est, depuis 1991, un véritable moteur du développement local. Il apporte un soutien à l'innovation, à la mise en réseau et à la coopération dans nos territoires ruraux. Nous savons tous combien la constitution d'un dossier pour demander des fonds Leader peut être fastidieuse et nous savons aussi combien le versement s'apparente à un véritable parcours du combattant au sein de l'enveloppe initiale de 700 millions d'euros, seuls 4 % auraient été versés ... Vous reconnaîtrez, monsieur le ministre, qu'il nous faut mieux faire ! Oui, je le reconnais ! À l'heure où l'on reproche trop souvent à l'Europe d'être éloignée de nos concitoyens, le programme Leader est un axe fort de son action au bénéfice des territoires ruraux. Il nous faut aussi mieux faire, parce que, derrière ces aides non versées, des artisans, des commerçants, des acteurs sociaux et culturels et de nombreuses communes sont fragilisés.

Alors que le président de Leader France parle de « crash généralisé » et que de trop nombreux projets sont à l'arrêt, pouvez-vous, monsieur le ministre, nous rassurer sur le versement des fonds prévus pour la période 2014-2020 avant son terme ? Enfin, ? Enfin, à l'heure de la négociation du cadre financier pluriannuel 2021-2027, pouvez-vous nous rassurer sur le maintien de l'enveloppe actuellement octroyée dans le cadre du dispositif Leader ? La parole

échelons décisionnels et en donnant davantage de pouvoirs aux régions. Celles-ci ont aujourd'hui une autorité de gestion. Donnons-leur aussi l'autorité en matière citoyen et écologiste. À la veille du 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, les femmes n'ont toujours pas obtenu l'égalité professionnelle qui passe par un salaire égal à celui des hommes pour un travail de valeur égale : elles perçoivent en moyenne 26 % en moins en France- faut-il encore le rappeler ? Pourtant, l'arsenal législatif existe pour parvenir à l'égalité professionnelle. Tout récemment, les mobilisations des femmes, des associations féministes et des organisations syndicales unies ont permis d'obtenir une avancée en matière d'égalité salariale avec la mise en place d'une obligation de résultat pour les entreprises. La ministre du travail, Muriel Pénicaud, y a contribué, comme elle s'y était engagée ici même lors l'examen du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Hélas, disposition après disposition, le décret vide de son efficacité le dispositif que nous avons adopté en juillet dernier. Pourquoi le Gouvernement a-t-il retenu des modalités de construction de l'index de l'égalité salariale qui permettent aux entreprises de dissimuler les écarts de rémunérations, allant ainsi à l'encontre du pouvoir législatif ?

Selon le, il faudrait, au rythme actuel, attendre 2234 pour obtenir une parité parfaite ... Nous refusons d'attendre deux siècles ! C'est pour cette raison que la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de septembre 2018 prévoit une obligation de résultat et une transparence des entreprises sur ces questions.

Il est assorti d'une sanction, qui peut aller jusqu'à 1 % de la masse salariale. En effet, les engagements pris par les entreprises ne doivent pas être en chocolat ! Il est également propice

En réalité, vous avez choisi des indicateurs qui rendent invisibles les discriminations et quasi inopérantes les sanctions, car vous les avez rendues de fait exceptionnelles. Pire, vous avez même introduit un seuil de tolérance de violation de la loi ! Les femmes qui manifestent dans la rue depuis des mois pour obtenir plus de pouvoir d'achat, en exigeant notamment une hausse des salaires et des minima sociaux, ne peuvent se satisfaire d'un tel tour de passe-passe, comme les organisations syndicales et les associations féministes qui dénoncent la précarité et le retour au temps partiel imposé et demandent la revalorisation des métiers à prédominance féminine. Je serai dans la rue à leurs côtés demain, à 15 heures 40, heure symbolique, pour dénoncer le travail gratuit effectué quotidiennement par les femmes. À l'heure où le Gouvernement cherche des financements et fait la poche des pauvres, l'égalité salariale

Mme la ministre du travail. La crise sociale profonde que traverse notre pays ces derniers mois jette une lumière crue sur l'ampleur et l'aggravation des inégalités dans notre société. Et il suffit d'observer les cortèges qui défilent dans nos rues pour constater que les femmes sont particulièrement frappées par cette précarité. En cette veille de 8 mars, Journée internationale des femmes, il est impossible de ne pas s'indigner du fait que l'égalité des chances, qui est tant recherchée, ne s'opère pas avec la même force, que l'on soit un homme ou une femme.

Si l'intention est louable, nous ne pouvons que regretter le manque d'ambition de cette mesure. Pourquoi la limiter aux grandes entreprises, quand plus de 48 % de l'emploi salarié se trouve dans les PME ? PME ? Surtout, comment croire en cet indicateur, si les entreprises s'évaluent elles-mêmes ? Je rappelle en outre qu'au 1 mars seule la moitié des entreprises s'est pliée à cette obligation ... L'indispensable lutte contre les inégalités ne peut se réduire à un tableau de chiffres. Elle doit passer par une politique volontariste et coercitive, sanctionnant les discriminations avec la plus grande sévérité. Nous ne pouvons plus accepter que, comme le démontre une étude publiée par le ministère du travail l'année dernière, 62 % des femmes aient connu ou connaîtront la précarité professionnelle au cours de leur carrière contre seulement 32 % des hommes. Alors que le Président de la République a déclaré que l'égalité entre les femmes et les hommes devait être une grande cause de son quinquennat, quelle est la réalité ? La vérité, c'est que le budget consacré à cette lutte ne représente que 80 millions d'euros, soit 0,0066 % du budget.

: congés de maternité, évolution des modes de garde des enfants, transparence dans l'attribution des places en crèche ... Cela passe également par l'entreprenariat au féminin

Le président Macron a affirmé au salon de l'agriculture que l'Europe doit avoir une politique agricole basée sur trois piliers forts : protéger, transformer et anticiper. Le groupe allemand Südzucker,

pas la moindre concertation ! Heureusement que la France et l'Allemagne sont étroitement unies par différents traités de coopération, le dernier ayant été signé à Aix-la-Chapelle ... Heureusement que la politique agricole commune existe depuis le traité de Rome. Qu'en serait-il autrement ? À la veille des élections européennes, ce capitalisme débridé n'illustre pas de façon positive la coopération, pourtant souvent vantée, entre nos deux pays. Cette décision, si elle devient effective, condamnera d'importants bassins de production de betteraves dans la Somme, l'Aisne, l'Oise et le Pas-de-Calais et affectera 1 275 exploitations agricoles, soit plus de 20 000 hectares. Tout l'écosystème local avec plus de 600 emplois directs et indirects est déstabilisé et remis en cause : les salariés de l'usine, les transporteurs, les sous-traitants, les commerces locaux et les entrepreneurs agricoles sont violemment affectés. Il est aujourd'hui impératif de préserver l'intégrité d'une filière française qui contribue chaque année pour 1,3 milliard d'euros à réduire le déficit de notre balance commerciale. Le Gouvernement doit tout mettre en oeuvre pour éviter cette décision, qui mettrait en danger une filière performante

elle avait fait l'objet d'un vrai travail de convergence, d'un vote à l'Assemblée de Corse et d'un décret. Elle permettait d'appréhender les perspectives énergétiques de la Corse, en misant sur une véritable politique d'efficacité énergétique une meilleure intégration des énergies renouvelables dans le énergétique, tout en prenant en compte la vétusté de certains moyens de production, comme la centrale du Vazzio, et l'interconnexion entre la Corse et l'Italie. aujourd'hui que cette PPE, unanimement saluée à l'échelon national comme localement, qui avait obtenu toutes les validations des différentes commissions nationales et qui avait réussi à emporter l'accord de la majorité des parties prenantes en Corse, semble être remise en question.

Madame la ministre, pourriez-vous nous faire connaître les intentions du Gouvernement concernant la prochaine PPE en Corse, notamment au regard des éléments majeurs présents dans l'actuelle programmation ? Vous devez savoir qu'il y a urgence et que les Corses n'accepteront jamais une prolongation des anciens moyens de production qui doivent normalement être déclassés en 2023,

de poursuivre un fonctionnement au fioul lourd, ce qui est inacceptable pour la population du pays ajaccien. Plus précisément, pouvez-vous nous dire, madame la ministre, si oui ou non le Gouvernement a l'intention de respecter le décret du 18 décembre 2015 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie en Corse, qui prévoyait la réalisation d'une infrastructure d'alimentation en gaz naturel de la Corse, la construction, avec un objectif de mise en service au plus tard début 2023, d'un cycle combiné d'une puissance de 250 et la conversion des moyens thermiques existants au gaz naturel. La parole

situées à Ajaccio et à Bastia, qui sont vieillissantes et polluantes. La PPE de 2015 a prévu que ces installations seraient remplacées par des centrales à gaz. À cet effet, un projet consistait à installer une barge de gaz à Bastia et à relier cette dernière par un gazoduc traversant la Corse pour alimenter la seconde centrale Les difficultés sont cependant très nombreuses, comme vous le savez, monsieur le sénateur, en particulier parce que le trajet du gazoduc doit passer non seulement au travers de la montagne, mais aussi au milieu de parcelles privées, dont le régime juridique est particulièrement complexe ... Le ministre

envisagé de nouvelles pistes, qui pourraient passer par l'installation d'un second terminal de gaz, potentiellement immergé en mer au large d'Ajaccio. Le Gouvernement est résolu à tenir ses engagements dans le cadre de la nouvelle PPE et entend bien évidemment s'assurer du renforcement de la sécurité énergétique de la Corse, tout en développant les énergies renouvelables. La parole est à Mme Annick Billon, pour le groupe Union Centriste. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Mme la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. En novembre 2017, le Président de la République annonçait vouloir faire de l'égalité entre les hommes et les femmes la grande cause nationale de son quinquennat. En cette veille de 8 mars, je souhaiterais évoquer la question alarmante des féminicides. Le nombre de femmes tuées augmente de façon inquiétante depuis le début de cette année. En effet, depuis janvier 2019, trente femmes ont été victimes de leur conjoint ou ex-conjoint. C'est deux fois plus que l'année précédente sur la même période. Elles sont plus de deux cents à avoir succombé ces deux dernières années. Plus généralement, environ 225 000 femmes sont victimes de violences conjugales, physiques ou sexuelles. En 2018, dans le sillage de l'affaire Weinstein, les plaintes pour viol ont augmenté de près de 17 % et celles pour agression sexuelle ont bondi d'environ 20 %. Or le nombre de condamnations effectives, lui, stagne. On le sait, la formation des personnels de police sur ces questions n'en est qu'à ses balbutiements. Par ailleurs, la délivrance d'ordonnances de protection par les juges aux affaires familiales, en principe accessibles à toutes les victimes de violences conjugales sans nécessité de dépôt de plainte préalable, est loin d'être systématique. La lutte contre les violences conjugales doit être appréhendée de manière globale en incluant les individus, les travailleurs sociaux, les magistrats, les forces de l'ordre et les associations. d'euros sur les 420 millions d'euros des crédits consacrés à l'égalité sont alloués chaque année à la lutte contre les violences faites aux femmes. Il faudrait cinq fois plus de moyens, car la mise en place de politiques publiques a un réel impact sur la hausse ou la baisse du nombre de victimes. À la veille de cette journée hautement symbolique, le Gouvernement se donne-t-il réellement les moyens de lutter contre les féminicides ? La parole

vouloir excuser l'absence de ma collègue Marlène Schiappa. Je vais répondre à sa place sur ce sujet de l'égalité entre les femmes et les hommes. Vous le savez, c'est la grande cause du quinquennat.

loi créant le délit d'outrage sexiste, permettant de verbaliser le harcèlement de rue. La France est le premier pays au monde à mettre en oeuvre cette mesure. Et cela fonctionne : en six mois, plus de 330 amendes, allant jusqu'à 750 euros, ont été infligées. Ce dispositif fera l'objet d'une évaluation parlementaire à partir du début de l'été, ce qui permettra de proposer d'éventuels correctifs. correctifs. Je pense aussi à la loi portée par Muriel Pénicaud sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Madame la sénatrice, vous m'interrogez sur les violences faites aux femmes et les féminicides. Nous nous sommes engagés très rapidement sur la création de centres de prise en charge du psychotraumatisme, notamment dédiés aux femmes victimes de violences, sexuelles ou autres, de la part de leur conjoint. Nous avons lancé un appel à projets et à candidatures l'année dernière ; dix centres ont été créés et labélisés. Notre pays est le premier au monde à organiser des réseaux de prise en charge des victimes

efficacement pour améliorer la desserte des territoires fragiles et victimes d'un enclavement mortifère, souvent à la fois routier, ferroviaire, aérien, et même numérique. Le Sénat a voté, le 20 février 2019, par 305 voix, la proposition de loi du RDSE relative à ce sujet capital pour ces territoires, et nous attendons avec espoir que la loi d'orientation des mobilités reprenne en grande partie ces propositions largement partagées. Un des sujets abordés par la proposition de loi est le transport aérien régional, en particulier les lignes d'aménagement du territoire. Certes, vous avez prévu un effort budgétaire, que nous saluons, mais, sur le terrain, force est de constater la qualité de plus en plus déplorable du service rendu aux usagers- annulations fréquentes, retards mettant parfois en jeu leur sécurité -, et ce en dépit du prix prohibitif des billets et du financement public État-collectivités. de constater le quasi-monopole d'une compagnie nationale pour laquelle ces liaisons sont malheureusement considérées comme secondaires, voire comme une charge. Il n'est pas concevable, en 2019, que nos compatriotes habitant dans ces territoires particulièrement fragiles soient traités de la sorte. Madame la ministre, je vous poserai deux questions simples.

quelles mesures entendez-vous mettre en place pour que les lignes aériennes d'aménagement du territoire permettent aux voyageurs de bénéficier d'un prix raisonnable et d'une qualité de service digne de ce nom ?

j'ai eu l'occasion de le dire lors de l'examen du texte, je partage largement les constats de la proposition de loi que vous avez évoquée, et la loi d'orientation sur les mobilités y répondra. Concernant les liaisons aériennes d'aménagement du territoire, je suis convaincue qu'elles sont essentielles pour nos territoires. C'est pour cette raison que j'ai souhaité relancer ces liaisons en quadruplant le budget qui leur est consacré. Dès 2019, l'augmentation de ce budget va se traduire par des améliorations concrètes à Limoges, Castres, Quimper, Poitiers et La Rochelle. Nous n'avons donc pas attendu pour agir. Au-delà de cet engagement de l'État, il est effectivement primordial de redresser la qualité de service de ces dessertes, et nous sommes fortement mobilisés pour ce faire. Voilà plusieurs mois, j'ai demandé un programme d'action à Hop !, qui a permis notamment de réduire le nombre d'incidents techniques et donc le nombre d'annulations. J'ai échangé avec le nouveau directeur général d'Air France-KLM et avec la nouvelle directrice générale d'Air France, qui sont pleinement conscients de la nécessité d'améliorer la qualité de service sur ces liaisons. Ainsi, l'organisation et la gestion des vols vont être reprises directement par Air France et les appareils de type ATR vont être retirés de la flotte en 2020. Au demeurant, ces liaisons sont remises régulièrement en concurrence, et on peut donc espérer que ce soit l'occasion d'améliorer la qualité de service. Je peux vous assurer, madame la sénatrice, que le Gouvernement est pleinement mobilisé sur

La parole est à Mme Laurence Harribey, pour le groupe socialiste et républicain. En 2017, le Gouvernement avait fait de la réindustrialisation une priorité, mais les faits sont cruels : 850 emplois rayés de la carte chez Ford, 450 emplois chez Ascoval suspendus à des plans de reprise, jeu à la Fonderie du Poitou, 900 sur les sites papetiers sarthois d'Arjowiggins. La liste n'est pas close. Le Gouvernement a trouvé indigne l'attitude de Ford et s'est dit trompé dans la reprise avortée d'Ascoval. Au-delà de l'indignation, quelle est la colonne vertébrale de la politique industrielle ? Pourquoi se désengager d'industries stratégiques, alors que d'autres font le contraire, des États-Unis à la Chine, en passant Sur ce point, les reproches faits aux Pays-Bas pour leur attitude envers Air France-KLM étonnent au regard de l'énergie déployée pour privatiser quelques fleurons profitables, par exemple Aéroports de Paris.

Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, madame la sénatrice Harribey, les faits sont têtus : la France

un peu de calme ! ... qui permet le développement de l'activité économique en rendant la plateforme française plus compétitive. C'est ce qui explique que Toyota investisse 300 millions d'euros en France, Daimler 500 millions d'euros, et que nous soyons désormais la première destination des investissements directs à l'étranger pour l'industrie. Nous poursuivons une politique industrielle de développement des contrats stratégiques de filière pour dix-huit filières, avec des projets d'innovation et de compétences. Quel est le premier point de blocage pour les emplois industriels ? C'est le recrutement, madame la sénatrice, qui empêche la croissance 50 000 emplois ne sont pas pourvus aujourd'hui dans l'industrie ! Si l'on était capable de mettre les compétences face aux chefs d'entreprise,

Permettez-nous de vous proposer quelques pistes de travail. Osons des prises de participation temporaires en cas de crise, comme l'a fait le président Obama pour General Motors ou la France, dans d'autres temps, pour Peugeot. Responsabilisons les grands groupes, donneurs d'ordre des PME : si Renault pérennise ses commandes à la Fonderie du Poitou, la reprise devient crédible.

qui a accompagné près de 300 entreprises, représentant 35 000 emplois, en deux ans. Osons la coopération industrielle européenne, à l'image d'Airbus, en étant porteurs d'une vision européenne. Voilà les pistes sur lesquelles nous sommes prêts à travailler ! La parole est La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le Premier ministre. Ah ! Le « prisonnières du hijab » fleurit sur les réseaux sociaux de l'autre côté de la Méditerranée. Derrière, il y a des femmes courageuses qui dénoncent le voile comme un instrument d'oppression. Elles pointent du doigt la pression sociale et l'environnement familial, qui les condamnent à se voiler. Chez nous aussi, la pression des quartiers et des familles ne laisse en réalité que peu de choix aux femmes voilées, en particulier aux plus jeunes d'entre elles. Alors que les femmes algériennes nous indiquent la voie du courage, la position de votre majorité est, sur ce sujet, d'une ambiguïté problématique. Or la France, nation des droits de l'homme, doit véhiculer un message de liberté pour les femmes du monde entier. Le Président de la République, le 16 avril 2018, déclarait que le voile n'était pas « conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays ». Le 28 février dernier, il se muait en défenseur du voile, expliquant que « les entreprises qui discriminent les femmes voilées à l'embauche [devaient être] sévèrement sanctionnées Sur ce sujet, l'exécutif fait donc preuve d'angélisme, pire, de contradiction ! Pouvez-vous, monsieur le Premier ministre, au nom du Gouvernement, devant notre assemblée, condamner de nouveau les propos d'un député de votre majorité qui a réalisé, la semaine dernière, un amalgame surréaliste entre le port du hijab et celui du serre-tête ? Alors que se célèbre demain la Journée de la femme, il est essentiel de rappeler que le combat pour une véritable égalité hommes-femmes passe aussi par le combat, sur notre territoire, contre toute forme de fondamentalisme, dont le voile est souvent un étendard. Monsieur le Premier ministre, le voile est-il, oui ou non, un instrument d'oppression des femmes ? Que comptez-vous faire pour protéger toutes ces femmes qui, sur le territoire français, sont contraintes de le porter ? La parole

je rappellerai simplement que nous sommes dans un pays où la laïcité est la règle ; elle s'inscrit au fronton de toutes nos mairies et de toutes nos institutions. Je crois que nous devons respecter également la volonté de chacun de porter ou non les attributs vestimentaires qu'il souhaite dans l'espace public.

afin que nous puissions partager nos convictions de façon universelle sur les violences faites aux femmes, sur les contraintes faites aux femmes, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'émancipation des femmes, autant de concepts, qui, à notre sens, doivent être universels, et qui nécessitent un engagement de toutes et tous,

que le Président de la République remettra le prix Simone-Veil, qui récompense les actions en faveur des droits des femmes dans le monde.

Madame la secrétaire d'État, je prends acte de votre réponse. J'ai bien peur qu'elle ne soit en total décalage avec le sens de mon message. Bien sûr ! Vous devez réaffirmer les valeurs d'universalisme qui font l'ADN de la France. Vous devez nommer les problèmes pour mieux les combattre. Le relativisme, qui est la marque de votre gouvernance depuis le départ, est une mauvaise réponse à de vrais problèmes. Je vous demande d'y réfléchir. Il est temps, vraiment

Pardonnez-moi si, en tant que sénateur de l'Orne, je n'ai pas exactement la même vision de la situation. Évidemment, je m'associe à la solidarité exprimée à l'égard des victimes de cet attentat, mais j'oscille entre colère et découragement. comprendre l'improbable et surréaliste régime des fouilles, alors que plus de 90 000 objets ont été trouvés cette année, et que 40 000 téléphones sont entrés dans les prisons en 2017

Comment expliquer également l'accès à une unité de vie familiale pour un criminel de cette nature, qui plus est deux fois par mois ? Comment expliquer les failles du renseignement pénitentiaire, alors que ce détenu était signalé pour des faits de radicalisation ?

votre réflexion sur la question de la radicalisation. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de lire ce que vous aviez écrit hier et avant-hier sur ce sujet. Je voudrais ici vous assurer que la détermination du Gouvernement pour lutter contre la radicalisation en prison est totale

Tout d'abord, nous avons agi pour prendre en charge ces personnes radicalisées. Vous me demandez un calendrier, je vous le donne. Depuis le mois de janvier dernier, nous avons développé des processus d'évaluation de la radicalisation. Ils sont en cours de déploiement. Nous avons aujourd'hui cinq quartiers d'évaluation de la radicalisation, là où il n'y en avait que deux l'année dernière. nous avons mis en place un système qui permet d'affecter ces détenus radicalisés dans des lieux adaptés. Ce sont des quartiers d'isolement ou ou des quartiers de prévention de la radicalisation, en tout état de cause des quartiers étanches du reste de la détention, pour éviter le prosélytisme. Mais cela se construit progressivement.

accru de plus de 16 % le budget de sécurité des établissements pénitentiaires. Là encore, nous allons continuer. Enfin, nous avons pris des mesures pour protéger nos personnels pénitentiaires. Ces mesures de protection, contrairement à ce que vous avez affirmé à l'instant, passent notamment

Plus de 1 500 gilets ont été déployés, et ce n'est pas terminé. D'autres mesures sont également prises dans ce sens. La sécurité des Français est notre priorité ; celle des personnels pénitentiaires l'est tout autant, madame la sénatrice.

années. Je voulais simplement indiquer que la radicalisation en prison ne date pas d'hier ; elle ne date pas non plus de votre gouvernement. Farhad Khosrokhavar l'a dénoncée depuis extrêmement longtemps. On sait qu'il faut laisser du temps au temps, et c'est normal, mais vous voyez bien que les personnels manquent quand même d'équipements. Ils manquent aussi de formation. Quant à l'évaluation, qui est un sujet

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour le groupe Les Républicains. messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, ministre de tutelle d'Atout France, organisme chargé de la promotion de la destination touristique France Il semble, en effet, qu'une note interne au Quai d'Orsay envisage un plan d'économies drastiques à Atout France, entraînant un plan social de grande ampleur. Celui-ci aura pour conséquence de réduire d'un tiers la masse salariale et d'économiser près de quatre millions d'euros. L'opérateur Business France serait aussi concerné. Évidemment, nous ne sommes pas contre de nécessaires économies dans l'usage des deniers publics, bien au contraire. convenez, monsieur le ministre, que cette coupe claire entraînerait la fermeture de plusieurs bureaux à l'étranger et impacterait grandement les missions de rayonnement et d'attractivité des destinations françaises, dont Atout France a la charge. Alors que notre pays subit depuis plusieurs semaines une dégradation de son image auprès des touristes étrangers en raison des mouvements sociaux de grande ampleur que nous subissons, monsieur le ministre, quelles sont vos ambitions pour la promotion du tourisme auprès des clientèles étrangères ?

le tourisme est un secteur clé pour notre économie, en même temps qu'un instrument d'influence majeure à l'étranger. C'est pourquoi le Gouvernement fait du développement touristique de l'ensemble des destinations françaises l'une de ses priorités. Les objectifs que nous nous sommes fixés en matière de fréquentation et de retombées économiques sur les prochaines années sont ambitieux. Les résultats de 2018 sont à cet égard encourageants, avec près de 90 millions de touristes étrangers, mais nous devons encore faire davantage, et Atout France est au coeur, évidemment, de cette stratégie. Vous évoquez la question des moyens. Les grandes orientations données par le Gouvernement dans le cadre d'Action publique 2022 impliqueront nécessairement, et c'est logique, une transformation de la présence internationale de l'État, de ses opérateurs, et donc d'Atout France, après évaluation de l'efficacité de l'action de chacun. Nous aurons donc très rapidement à mener une réflexion stratégique stratégique sur la meilleure manière d'assurer la promotion touristique de nos destinations à l'étranger avec Atout France et ses partenaires publics et privés. En ce qui concerne plus particulièrement le financement de la promotion touristique, le Gouvernement s'est clairement engagé, lors du conseil interministériel du tourisme du 19 janvier 2018, en apportant des ressources supplémentaires pérennes, notamment par le biais de la recette « visas Le ministre Jean-Yves Le Drian et le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne resteront mobilisés pour que les collectivités, les professionnels et l'État rassemblent leurs énergies et leurs moyens en faveur de la promotion des destinations, dans un modèle partenarial qui caractérise notre politique touristique et qu'incarne Le Gouvernement a également conforté Atout France dans sa mission d'appui à la structuration de nos offres touristiques. C'est le sens de la mise en place du dispositif France tourisme ingénierie, porté par Atout France et la Banque des territoires, qui accompagne les collectivités locales dans la structuration de projets touristiques d'envergure à même de répondre à une demande mondiale toujours plus exigeante. C'est en agissant à la fois sur la demande et sur l'offre que nous pourrons atteindre nos objectifs de fréquentation et de recettes touristiques. En affirmant plus encore la vocation touristique de notre pays,

Madame la ministre, après un début de quinquennat exécuté à marche forcée, nous constatons tous un net ralentissement de la marche. Depuis le 15 janvier, le temps législatif est figé et on ne compte plus les projets de loi reportés et les réformes suspendues aux conclusions du grand débat national. Plus grave encore, sans doute, le travail parlementaire est désormais balayé d'un revers de manche par votre gouvernement. Ainsi, le 11 décembre dernier, le Sénat votait à une très large majorité une proposition de loi, déposée par notre collègue Françoise Gatel et rapportée par Agnès Canayer, qui visait

vous avez rappelé l'importance des communes nouvelles, qui ont été créées par la loi de 2010 et réformées en 2015 par le député Jacques Pélissard. Cette politique est un grand succès puisque, aujourd'hui, 2 508 communes se sont regroupées pour créer 774 communes nouvelles. On peut s'en féliciter, ne serait-ce que parce qu'il y en a encore eu 239 En conséquence, le nombre de communes est aujourd'hui de 34 970, pour être très précise. On le sait, monsieur le sénateur, cette politique a beaucoup de succès, particulièrement dans l'ouest de la France, notamment dans le département de Maine-et-Loire que vous représentez ici au Sénat, mais aussi dans la Manche,

La proposition de loi, adoptée par la Haute Assemblée en décembre dernier, vise en ce sens à faciliter le développement des communes nouvelles et à améliorer, surtout, les périodes transitoires, notamment pour ce qui concerne la composition des conseils municipaux, la deuxième période. Ce texte a été reçu très positivement. Il a été soutenu par le Gouvernement. Aujourd'hui, il est bien sûr nécessaire d'envisager sa lecture,

voir le mal quelque part mais, aujourd'hui, c'est le Gouvernement qui bloque, qui ne veut pas comprendre qu'il y a urgence à légiférer sur ce texte, notamment à l'approche des futures élections municipales. J'entends bien votre volonté affichée d'être à l'écoute, et je m'en félicite- c'est un changement notable. Peut-être pourriez-vous aller jusqu'à entendre la volonté des parlementaires qui travaillent et se saisissent des attentes des élus locaux, en étroite collaboration d'ailleurs avec l'Association des maires de France ? Peut-être pourriez-vous, collectivement, au sein du Gouvernement, consacrer un peu moins de temps à l'animation du médiatique de votre mentor

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, il y a quelques années, en février 2014, notre collègue Mireille Schurch présentait ici même une proposition de loi du groupe CRC permettant d'engager la renationalisation des concessions autoroutières. L'ensemble des groupes siégeant sur ces travées, à l'exception des communistes et des écologistes, avaient alors rejeté ce texte, préférant reporter l'examen de cette question et attendre la fin des concessions, comme l'y invitait, d'ailleurs, le Gouvernement. Cette position s'est révélée non seulement hasardeuse, mais également peu pertinente, car la fin des concessions n'a depuis lors cessé de s'éloigner. En effet, en s'engageant dans un cycle de renégociation particulièrement opaque dès 2015, le Gouvernement a, au final, fait perdurer un système défavorable aux intérêts publics, un protocole tellement insatisfaisant qu'il oeuvre depuis lors pour en cacher le contenu malgré les assignations en justice. Nous rouvrons donc, cinq cinq années plus tard, le même débat avec la même proposition de loi, en espérant que la prise de conscience autour de ce scandale d'État aura continué de faire son chemin. Ces derniers mois ont d'ailleurs démontré que les questions de maîtrise publique des infrastructures revenaient avec force, que ce soit dans nos débats parlementaires, autour de la privatisation d'Aéroports de Paris, ADP, que le Sénat a rejetée, tout autant que dans la rue et sur les ronds-points au travers du mouvement des « gilets jaunes », qui ont fait de la renationalisation des autoroutes l'une de leurs propositions structurantes, notamment la plateforme de revendication mise en ligne en novembre dernier. Le fait que ces mouvements aient organisé des initiatives « péages gratuits » n'est pas non plus anodin, les autoroutes étant devenues l'un des symboles d'un racket organisé sur des usagers captifs avec la complicité/passivité du Gouvernement. Il faut dire que la colère est légitime : la rente des sociétés concessionnaires a cela de scandaleux qu'elle illustre parfaitement la captation d'un bien public au profit d'intérêts privés. d'une véritable spoliation puisque ces infrastructures ont été financées par l'impôt de tous. Il me semble aujourd'hui- et c'est déjà un progrès -que le constat est partagé quasi unanimement concernant l'erreur que fut la vente des autoroutes en 2006 par le gouvernement Villepin, une décision prise dans la précipitation, guidée par la seule obsession de réduire le déficit public. Je ne reviendrai donc pas sur les avis des différentes autorités, telles que la Cour des comptes ou l'Autorité de la concurrence, qui ont dénoncé cette situation. L'avis de l'Autorité de la concurrence avait très bien résumé la situation : elle mettait ainsi en évidence la « rentabilité exceptionnelle » de ces sociétés, une rentabilité qui n'est pas justifiée par les risques ou les coûts supportés par ces sociétés. Une telle constatation nous conduit d'ailleurs à penser, comme cela est suggéré par certains juristes, que l'on pourrait précisément remettre en cause les concessions autoroutières- du moins pour les concessionnaires historiques -sur ce fondement, en faisant de l'absence d'aléa dans la prise de risque un vice permettant de les dénoncer. En effet, le Conseil d'État a déjà estimé que l'une des parties à un contrat administratif pouvait en obtenir la mise à l'écart lorsque ce contrat est entaché « d'un vice d'une particulière gravité relatif aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement une piste que personne n'a pour l'instant voulu suivre. Aujourd'hui, il devient pourtant urgent de mettre un terme à cette situation, qui pèse non seulement sur les comptes publics puisque cette privatisation a privé l'État d'une manne financière de 32 milliards d'euros, mais également sur les usagers, considérés comme de simples réservoirs à dividendes pour les actionnaires. Actuellement, les sociétés d'autoroutes françaises se portent plutôt bien, avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 8 milliards d'euros, d'euros, en augmentation de 42,3 % entre 2009 et 2016, d'après le Commissariat général au développement durable, le CGDD. Ces sociétés font dans le même temps des bénéfices record, 4,7 milliards d'euros de dividendes pour l'année 2016, selon l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Arafer. Grâce à ces bénéfices, les sept sociétés ont déjà remboursé ce qu'elles avaient mis sur la table pour acheter les parts de l'État : 14,8 milliards d'euros. selon les chiffres de l'Arafer, l'ensemble des sociétés autoroutières a dégagé un excédent brut d'exploitation de 7,3 milliards d'euros pour 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une marge brute de 73 %. Certaines sociétés concessionnaires n'hésitent pas non plus à emprunter pour verser des dividendes. Dans le même temps, les tarifs ont augmenté de 20 % environ en dix ans. Face à cette situation et à l'émotion populaire suscitée, le Gouvernement avait engagé dès 2014 une réflexion, qui s'est traduite par la renégociation des concessions et la signature d'un protocole d'accord. Un gel des tarifs a ainsi été décidé en 2015, mais la hausse sera simplement reportée sur les années 2019 à 2023. Chaque plan autoroutier adopté par l'exécutif gouvernemental a, par ailleurs, et contre toute attente, défini un allongement de la durée des concessions. Le protocole d'accord, signé le 9 avril 2015 par les ministres Ségolène Royal et Emmanuel Macron, prévoit ainsi que les 3,2 milliards d'euros d'investissements financés par les sociétés d'autoroutes seront compensés par une prolongation de la durée des concessions de deux ans et demi en moyenne, certaines concessions étant même prolongées de cinq années. En 2017, des avenants ont été signés. Ils prévoyaient 800 millions d'euros d'investissements sur le réseau moyennant une hausse de 0,4 % des péages entre 2018 et 2020 et une participation des collectivités territoriales. Sur ces avenants, les conclusions de l'Arafer étaient particulièrement éloquentes. En effet, selon cette autorité chargée de la régulation du secteur, « il n'apparaît pas justifié de faire supporter par l'usager de l'autoroute le financement de vingt-trois Elle indiquait par ailleurs que « les augmentations de tarifs de péages prévues excèdent le juste niveau qu'il serait légitime de faire supporter aux usagers ». Pourtant, malgré toutes ces alertes, les tarifs ont encore augmenté au 1 février de 1,9 % en moyenne. Comment l'État peut-il rester indifférent à ce racket ? L'intérêt général est bafoué. Nous sommes face à une situation extraordinaire où des inquiétudes se font même jour sur l'incapacité de l'État à défendre ses intérêts et l'intérêt général face au privé. Depuis plus d'une décennie, les pouvoirs publics ont systématiquement fait les mauvais choix. pour sortir de ce piège et trouver la solution, il faut absolument poser le bon diagnostic sur les rapports de forces. Dans ce cadre, il faut bien se dire que les pratiques des sociétés concessionnaires sont absolument légales puisqu'elles découlent des contrats de concession signés par l'État. En effet, les contrats liant les concessions autoroutières à l'État sont aujourd'hui tellement bien ficelés que l'État reste pieds et mains liés, perdant et incapable d'imposer tout encadrement ou toute révision de ces contrats. Lorsque l'État demande une réduction des abonnements, c'est non pas une exigence fondée sur l'intérêt général, mais une simple aumône face à des sociétés qui se croient dans leur bon droit et sont ultrapuissantes. Comment s'en satisfaire ? C'est donc bien l'État lui-même qui a organisé volontairement sa propre défaillance et sa capitulation devant les intérêts des géants du BTP. Toute disposition qui pourrait changer les termes des contrats doit aujourd'hui donner lieu à compensation, selon les termes de l'accord, afin « d'assurer, dans le respect du service public, les conditions économiques et financières » des contrats- entendons un niveau de rentabilité extrêmement élevé. En gros, toute charge nouvelle sera compensée sur les usagers, ce qui n'est pas une option. Dans ce contexte, une seule solution existe. L'État a la possibilité, pour un motif d'intérêt général, comme cela est prévu à l'article 38 de chacun des contrats de concession, d'y mettre fin.

Au regard des taux d'intérêt actuels, le recours à l'emprunt semble une bonne option., cet argent emprunté sera remboursé non pas par l'impôt, mais par le péage. Nous pensons, par ailleurs, que l'État pourrait se mettre dans une position offensive et s'appuyer sur le principe constitutionnel interdisant aux personnes publiques de consentir des libéralités. Il est ainsi interdit à une personne publique de verser une indemnisation manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi, y compris à la suite d'une rupture anticipée d'un contrat administratif. Nous estimons que nous sommes tout à fait dans ce cas de figure, madame la ministre, au regard notamment de la sous-estimation initiale qui a lésé l'État dans la protection de ses intérêts. Encore une fois, nous pensons qu'il conviendrait que l'État mène cette bataille. Au moment où il existe une fronde légitime dans notre pays sur les taxes et la vie chère, cette option semble aujourd'hui plus que pertinente. Pour preuve de sa faisabilité, l'Espagne s'est engagée dans cette voie en annonçant la renationalisation de 500 kilomètres de tronçons, qui vont ainsi repasser sous maîtrise publique.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, politique. Avec cette proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes et à l'affectation des dividendes à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable a bien voulu me confier le rapport. Je salue au passage notre ancienne collègue Évelyne Didier, qui avait travaillé sur un texte similaire en 2014. Ce texte, qui a été déposé le 16 janvier dernier par notre collègue Éliane Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, vise à corriger l'erreur historique du gouvernement Villepin de 2006 et répond à une double actualité : premièrement, le renchérissement du coût de la mobilité pour nos concitoyens et la diminution de l'offre de transports collectifs, vivement soulignés par le mouvement des « gilets jaunes » et, deuxièmement, la privatisation d'Aéroports de Paris souhaitée par le Gouvernement, qui, comme celle des autoroutes, est symptomatique d'une politique de court terme où l'on dilapide les biens de l'État pour dégager des liquidités. Et j'ai la faiblesse de penser que, si la majorité sénatoriale s'est massivement opposée à la privatisation d'ADP, c'est qu'elle a pris toute la mesure du catastrophique précédent de la privatisation de 2006.

Pour mémoire, en 2019, le produit de cet impôt devrait dépasser 31 milliards d'euros. Précisons tout de même qu'il s'agit d'un gage pour les besoins de la procédure législative et que, naturellement, l'État n'aura aucune difficulté à faire l'avance de cette somme et à se rembourser les recettes des péages. C'est d'ailleurs ce que les sociétés d'autoroutes ont fait en 2006. En effet- c'est important de le rappeler -, nationalisation n'est pas synonyme de gratuité. Je vous présenterai donc, dans un premier temps, la position retenue par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, avant de vous faire part de trois remarques générales, que je juge utiles pour éclairer nos débats. Lors de sa réunion du 20 février dernier, la commission a souligné l'importance du sujet, en particulier dans le contexte social actuel, et la nécessité pour l'État d'user de l'ensemble des outils juridiques dont il dispose dont il dispose pour mieux réguler les concessions autoroutières et l'évolution des tarifs des péages supportés par les usagers. La commission a toutefois rappelé que la hausse importante des tarifs des péages constatée au 1 février 2019 est le fruit de décisions irresponsables prises par le passé.

Les différentes interventions des commissaires lors de l'examen de la proposition de loi ont ainsi permis de rappeler qu'un groupe de travail avait été constitué sur le sujet, en 2014, sur l'initiative de la commission. Coprésidé par MM. Jean-Jacques Filleul et Louis-Jean de Nicolaÿ, ce groupe avait notamment suggéré d'« avancer sur le chemin d'une reprise en main par l'État des concessions autoroutières », de façon progressive et si les circonstances le justifiaient, plutôt que d'envisager la piste d'un rachat généralisé des concessions, que certains avaient évoquée, Depuis 2014, les travaux menés par le Parlement et le Gouvernement ont abouti à un renforcement du dispositif législatif de contrôle des sociétés d'autoroutes. Les dispositions adoptées à cette fin dans le cadre de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont désormais inscrites dans le code de la voirie routière. La transparence de la régulation du réseau autoroutier concédé demeure toutefois largement perfectible ; à titre d'illustration, la commission n'a toujours pas pu avoir accès au protocole d'accord conclu en 2015 sous la houlette de Ségolène Royal et d'Emmanuel Macron. a conduit, entre autres choses, à un allongement jusqu'en 2036 de la durée des concessions, en échange de nouveaux travaux mis à la charge des concessionnaires, dans le cadre d'un plan de relance autoroutier de 3,27 milliards d'euros. Le ministère des finances refuse toujours de communiquer ce document, s'abritant derrière son « caractère transactionnel ». La question de la communicabilité de ce protocole sera tranchée la semaine prochaine par le Conseil d'État, à la suite des démarches d'un citoyen exigeant, Sans préjuger de sa décision, on se contentera de souligner que, le 20 février dernier, la rapporteure publique du Conseil d'État a conclu au rejet du pourvoi du ministre de l'économie d'alors, M. Emmanuel Macron, et à la communication de l'accord du 9 avril 2015 à M. Avrillier. Lors des auditions que j'ai conduites en tant que rapporteur de ce texte, j'ai renouvelé cette demande ; le même refus m'a été malheureusement opposé. C'est, à mes yeux, inacceptable, car il s'agit bien de l'argent du contribuable ! Aussi, je souhaiterais que Mme la ministre nous indique officiellement les raisons qui l'empêchent de transmettre ce protocole, pourtant essentiel au travail de contrôle de l'action du Gouvernement qui est confié au Parlement aux termes de la Constitution. Compte tenu du coût d'une renationalisation immédiate, sans doute supérieur à 50 milliards d'euros, de l'impréparation de l'État pour la reprise en main de l'exploitation des autoroutes, et de la proximité des échéances prévues pour certaines concessions, la commission a considéré, contre mon avis, que l'option de la renationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes devait être écartée. J'en viens maintenant aux trois remarques évoquées en introduction, qui sont essentielles pour la clarté de nos débats. En premier lieu, je considère que l'État s'est lié les mains avec la privatisation, s'enferrant toujours plus dans des montages contractuels complexes. Ainsi, en dépit des mauvaises expériences passées, l'État s'est réengagé en 2017 dans un plan d'investissement autoroutier. plan devait, à l'origine, s'élever à 900 millions d'euros, mais l'Arafer a réduit cette somme à 700 millions d'euros. Aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de défendre ni ses intérêts patrimoniaux ni l'intérêt général, en dehors d'un cadre contractuel qui a à peine évolué depuis le début de la construction des autoroutes, en 1955 deuxième remarque : à mon sens, l'exploitation des autoroutes n'est pas un marché risqué, même si la définition juridique d'une concession implique le contraire. Les bénéfices réalisés par les sociétés concessionnaires le confirment

En outre, la baisse des taux d'intérêt constatée depuis plusieurs années et soutenue par la politique accommodante de la Banque centrale européenne permet aux sociétés d'autoroutes de se refinancer à des taux bien plus faibles et donc avantageux. Enfin, les tarifs kilométriques moyens ont constamment augmenté, au-delà même de la formule d'évolution tarifaire annuelle fixée à 70 % de l'inflation, pour les sections historiques, et à 85 %, pour les sections récentes.

à un contrat d'objectifs et de performance comportant des critères forts en matière d'aménagement du territoire, d'efficacité environnementale et de différenciation des tarifs selon des motifs sociaux. Une telle idée me semble plus que pertinente. Ainsi, la fin des concessions permettrait d'avoir des débats sur la gratuité des autoroutes, la mobilité partagée, ou encore la mobilité connectée. Enfin, mes chers collègues, je vous rappelle qu'attendre la fin des concessions ne nous donne aucune garantie quant à de futures hausses de tarifs, du fait des nouveaux investissements qui pourraient être demandés par l'État aux sociétés concessionnaires. C'est un pari risqué ! C'est pourquoi le groupe CRCE et, à titre personnel, votre rapporteur proposent de renationaliser les sociétés concessionnaires d'autoroutes. La commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ne nous a toutefois pas suivis et a voté contre le texte. La parole

Monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, je sais que le sujet des concessions d'autoroutes intéresse beaucoup les parlementaires et nos concitoyens ; je suis donc ravie de pouvoir échanger avec vous sur ce thème. Concernant le coeur de cette proposition de loi- nationaliser les autoroutes en rachetant les sociétés concessionnaires -, je crois sincèrement que cette option n'est ni envisageable ni souhaitable.

sénateurs, je vous rappelle que, quand la concession arrive à échéance, le concessionnaire doit restituer l'ouvrage en parfait état. Les premières concessions arrivent à échéance en 2031. À l'échelle des durées des concessions, cette date est très proche. L'État n'a donc que peu d'intérêt à racheter à un prix exorbitant des concessions dont il commencera à retrouver la pleine propriété dans une dizaine d'années. Le Gouvernement est donc, vous l'aurez compris, défavorable à cette proposition de loi. En revanche, deux sujets méritent d'être évoqués : la relation entre l'État et les sociétés d'autoroutes, et la préparation de la fin des concessions. On pourrait dire beaucoup de choses sur les relations entre l'État et les sociétés d'autoroutes ; je commencerai mon propos par un rappel historique et des considérations générales. C'est la loi du 18 avril 1955 qui a autorisé l'État à créer des sociétés concessionnaires pour la construction et l'exploitation d'infrastructures autoroutières. Ces concessions, il faut le dire, ont permis de développer un réseau de routes très performant à un rythme qui n'aurait probablement pas été possible autrement. N'oublions pas que nous disposons, en France, d'un réseau autoroutier de plus de 9 000 kilomètres de voies concédées Je rappelle que ces sociétés étaient, au départ, pour l'essentiel publiques. Leurs bénéfices permettaient de financer les investissements dans les transports. Les concessions étaient alors à durée déterminée. Puis on a largement fait appel à l'adossement, notamment afin de financer le développement de liaisons interurbaines moins rentables.

elles servaient essentiellement aux trajets occasionnels des particuliers et au transport de marchandises sur de longues distances. Or, du fait de l'extension des agglomérations et des changements des modes de vie, on constate que beaucoup de Français sont aujourd'hui amenés à utiliser l'autoroute pour leurs déplacements quotidiens. Cela pose notamment la question de l'acceptabilité de ce modèle d'autoroute à péage pour ce type de trajets. Dans le même temps, le modèle d'une infrastructure financée entièrement par l'usager a un avantage dans un contexte où l'acceptabilité de l'impôt est, elle aussi, Parlons à présent de la privatisation des sociétés d'autoroutes survenue en 2005. Cette décision conduisait, par nature, à priver l'État des dividendes qui étaient jusque-là affectés aux investissements dans les infrastructures de transport. On peut s'étonner que cette évolution fondamentale n'ait pas été précédée de la révision de contrats qui, contrairement à ce que l'on observe généralement pour ce qu'on appelle les « actifs régulés » et notamment, en France, pour les aéroports, ne font pas l'objet d'un recalage périodique entre l'autorité concédante et le concessionnaire. Ces contrats conclus entre l'État et des sociétés d'économie mixte qu'il contrôlait alors régissent désormais ses relations avec des sociétés cotées, dont la logique est nécessairement différente. Je crois que le déséquilibre dans les relations entre l'État et les concessionnaires d'autoroutes vient de là ; cela explique les questions récurrentes sur les relations entre l'État et les concessionnaires. Cela dit, ce modèle a tout de même évolué, en particulier par l'accroissement de sa transparence à la suite, notamment, des travaux de l'Autorité de la concurrence. S'agissant de la transparence des relations contractuelles entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes, il convient de rappeler que la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

rend des avis publics sur les projets de nouveaux contrats de concession, mais aussi sur tous les projets d'avenants ayant une incidence sur les tarifs de péage. La Commission européenne, quant à elle, contrôle les renégociations de contrats ayant pour objet l'allongement de la concession, afin de s'assurer du respect du droit communautaire de la concurrence et de la commande publique. Le Parlement a également vu ses moyens de contrôle, d'évaluation et d'information considérablement renforcés. Depuis l'intervention qu'a représentée la loi du 6 août 2015 précitée, c'est ainsi au législateur qu'il revient d'autoriser l'allongement de la durée des contrats de concession. Par ailleurs, depuis 2009, le Parlement est chaque année destinataire d'un rapport sur l'exécution et le contrôle des contrats de concession d'autoroutes et d'ouvrages d'art, mais aussi d'un rapport sur l'évolution des péages pour chaque exploitant autoroutier. autoroutier. Il convient de souligner que, à la suite de la crise de 2015, s'est opéré un rééquilibrage des relations entre l'État et les sociétés concessionnaires. En effet, un dispositif limitant les surprofits a été introduit, autant que c'était possible, possible, dans les contrats historiques : en cas de surperformance économique sur la période d'allongement du contrat, les tarifs de péages sont revus à la baisse, ou la durée de la concession est réduite. L'État peut également récupérer l'avantage financier résultant des décalages constatés dans l'échéancier réel des investissements liés aux nouvelles opérations au regard de l'échéancier d'investissements contractualisé. Par ailleurs, des mécanismes d'incitation à la performance sont désormais prévus. Une liste d'indicateurs a notamment été établie : leur non-respect par les sociétés concessionnaires donne lieu à l'application de pénalités financières. Enfin, la loi du 6 août 2015 a créé l'Arafer, qui dispose d'un pouvoir de contrôle et de sanction de l'activité des concessionnaires. Ces éléments ont conduit, ces dernières années, à un certain rééquilibrage des relations entre l'État et les concessionnaires d'autoroutes. S'agissant S'agissant du protocole de 2015, monsieur le rapporteur, je crois que vous avez vous-même répondu à votre question relative à la communicabilité de ce protocole transactionnel : elle sera prochainement tranchée par le Conseil d'État. Au demeurant, les dispositions que ce

Je voudrais conclure sur ce point : demander aux sociétés concessionnaires de prendre leurs responsabilités était la seule voie. En effet, du fait des conditions de la privatisation que j'ai évoquée, l'État ne peut ni modifier l'équilibre du contrat avant son terme ni en changer la nature sans compensation. Je l'ai déjà dit : racheter les concessions ne me semble pas être une option. La priorité était de rééquilibrer les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires.

Si le choix de nouvelles concessions doit être fait, il faudra alors veiller à ce que les contrats soient équilibrés. L'État pourrait aussi bien évidemment choisir de gérer lui-même son réseau autoroutier. La situation actuelle n'est pas idéale, mais je crois qu'il faut tout faire pour l'améliorer et, surtout, penser à l'avenir. En tout cas, ce n'est pas en rachetant aujourd'hui les concessions que le financement de nos transports et l'entretien de nos infrastructures se porteront mieux. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je n'aurai pas recours à la facilité qui consiste à considérer le Premier ministre d'alors comme seul responsable de la situation qui est évoquée devant notre assemblée Pour autant, il nous faut bien reconnaître que, si les gouvernements successifs ont eu à coeur d'améliorer la performance de l'achat public,

ne manquait alors pas moins de 10 milliards d'euros pour que cette opération puisse être considérée comme ayant été réalisée au juste prix. De plus, les conditions dans lesquelles cette privatisation s'est opérée n'ont pas permis d'éviter que se constitue ce que d'aucuns qualifient- je ne suis pas loin de le penser également -de « rente » pour les sociétés concernées. Pire encore, ces dernières ont été incapables de protéger les intérêts légitimes des usagers, dont on sait que le recours à ces infrastructures s'est fortement accru ces dernières années. Ces rentrées d'argent vous auraient sans doute été très utiles, madame la ministre, à l'heure où vous défendez l'objectif d'une grande politique d'infrastructures et de mobilités.

il ne rend que d'autant plus ardues, voire hypothétiques, les chances de faire aboutir une nouvelle fois cette proposition.

que toutes les pistes visant à améliorer les recettes de celui-ci sont en proie à une contestation de plus en plus grande de la part de nos concitoyens, que l'État soit en mesure de mobiliser les 45 milliards d'euros nécessaires à l'aboutissement néanmoins souhaitable de cette Madame la ministre, nous sommes les représentants des territoires : celles et ceux qui nous élisent sont rompus à l'exercice des mandats locaux. Chaque année, ils font adopter un budget équilibré et sincère, comme l'exige la loi. Chaque année, dans la conduite des politiques publiques dont ils ont la charge, il leur arrive de procéder à des délégations de service public,

Cela devrait inspirer le gouvernement auquel vous appartenez, à l'heure où il propose la privatisation d'Aéroports de Paris. Si nulle économie collectiviste n'a fait la démonstration qu'elle était de nature à accompagner le développement personnel et collectif d'un pays, l'économie libérale, voire néolibérale, est tout aussi indigente ! Peut-être les excès de l'une et de l'autre permettront-ils de tirer les enseignements qui nous amèneront à légiférer différemment à l'avenir. À l'heure du grand débat il ne m'apparaît pas saugrenu de définir avec précision les politiques stratégiques qui ne peuvent ni ne doivent échapper au contrôle de la puissance publique, c'est-à-dire de la Nation tout entière, par le biais de ses représentants. Vous le voyez, mes chers collègues : bien que nous soyons conscients de la pertinence de la question posée au travers de cette proposition de loi, les conditions dans lesquelles la privatisation s'est opérée,

il nous apparaît impératif que l'État conserve les ingénieries administratives, juridiques et financières nécessaires pour que nous puissions mettre à profit la décennie qui nous sépare du terme des concessions de préparer au mieux le retour à une gestion par l'État de ces grandes infrastructures. Si, d'aventure, les données économiques s'amélioraient dans de telles proportions qu'il nous soit possible d'anticiper 2031,

À l'évidence, il serait malhonnête de ne pas reconnaître que les services de l'État n'ont pas été assez pugnaces lorsqu'il a été décidé, il y a maintenant près d'une vingtaine d'années, Concédé pour près de 15 milliards d'euros, le réseau autoroutier aurait en effet pu être mieux valorisé auprès des prestataires privés : à hauteur de 25 milliards d'euros, selon le rapport le plus récent de la Cour des comptes. Cour des comptes. Oui, l'objectif initial du Gouvernement, à savoir l'assainissement des comptes publics, n'aurait dû être que secondaire dans ses négociations avec les prestataires, au regard du creusement considérable du déficit et de l'alourdissement de la dette. À ce titre, il aurait mieux valu se concentrer sur la notion de service, en négociant des cahiers des charges plus exigeants et plus transparents. C'est d'ailleurs ce manque qui a longtemps constitué l'un des principaux reproches faits au système des concessions en matière autoroutière. Source régulière de débats, l'encadrement de l'augmentation des tarifs aurait également gagné à être beaucoup plus clair et transparent, conformément aux recommandations les plus récentes effectuées par l'Arafer.

Certes, le système de concessions aura fonctionné pendant près de vingt-cinq ans, mais la gestion et l'exploitation du réseau reviendront dans le giron de l'État dans une dizaine d'années. Charge reviendra alors aux pouvoirs publics de montrer qu'ils pourront faire mieux et moins cher sur ce sujet, ... Ce n'est pas difficile ! ... ce qui n'a rien d'une évidence pour le moment.

En outre, la rupture anticipée des contrats de concession entraînerait automatiquement une indemnisation des sociétés concernées et un alourdissement considérable de la dette publique. N'oublions pas non plus les 30 milliards d'euros de dettes portées en propre par les sociétés concessionnaires, que l'État devra donc logiquement reprendre à son compte. Enfin, en dépit de son intitulé, la proposition de loi ne comporte aucune disposition normative permettant d'affecter le produit des dividendes à l'Afitf. Il faut également rappeler une réalité concrète malgré tous les débats que nous pouvons avoir sur l'opportunité du recours aux concessions, le réseau autoroutier français, qui dépasse les 9 000 kilomètres, compte aujourd'hui encore parmi les meilleurs et les plus performants d'Europe. Citons à ce titre le rapport remis en 2017 par notre collègue Hervé Maurey, qui rappelait que 65 % du réseau était en très bon état, et près de 20 % en bon état. Cela correspond à un standard très exigeant dont peu d'États européens peuvent se targuer. Quant au fait que les concessions soient principalement détenues par de grands groupes, rappelons que rares sont les entreprises bénéficiant de la robustesse nécessaire pour assurer le fonctionnement d'un réseau aussi important. Bien entendu, cela ne signifie absolument pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et qu'il ne faut rien changer. Au contraire, il y a énormément de choses que nous pouvons faire à ce sujet. Nous pouvons améliorer la cohérence et la coopération entre les services de l'État et, notamment, entre le ministère des transports et Bercy, afin d'offrir une meilleure position à ces services lorsqu'ils négocient les contrats avec les concessionnaires. Nous pouvons exiger un meilleur usage des outils coercitifs dont dispose l'administration lorsque des manquements sont constatés tous les contrats comportent des clauses permettant à l'État de récupérer l'avantage financier découlant du retard d'une opération déjà compensée par des hausses de tarifs aux péages. Nous pouvons également améliorer la transparence de ces mêmes hausses de tarifs, dont il faut rappeler qu'elles sont annuellement encadrées par l'administration, et les ajuster en conséquence. Nous nous devons également d'être intraitables quant aux investissements en faveur de la modernisation des infrastructures, en nous assurant que ces derniers sont correctement évalués et effectivement mis en oeuvre. En revanche, nous ne pensons pas que la nationalisation permettra de régler à ce stade ces différentes problématiques. Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE, dans sa majorité, votera contre l'adoption de cette proposition de loi. La parole

La nationalisation des concessions autoroutières, qui s'accompagne, en filigrane, de la question des tarifs et du niveau des bénéfices des sociétés autoroutières, est certes d'actualité, mais elle représente également un fil rouge polémique depuis 2006. À titre d'exemple, nous avons encore en mémoire la tentative très médiatique, en 2014, de Ségolène Royal, qui envisageait la possibilité d'une résiliation des contrats de concession, en se fondant sur un rapport à charge de l'Autorité de la concurrence. La ministre avait très vite déchanté, car, selon les experts et le Gouvernement, une éventuelle renationalisation du réseau autoroutier aurait coûté- et coûterait même encore -50 milliards d'euros à l'État, lequel, soyons francs- comme vous l'avez rappelé, madame la ministre -, n'en a absolument pas les moyens. Une reprise paraît donc impossible. Le sujet de la gratuité des autoroutes fait également l'objet de vives discussions, notamment dans le cadre du grand débat national en cours. Cependant, même en faisant l'hypothèse que l'État dénonce les contrats passés avec les sociétés autoroutières, il semble évident qu'il serait obligé de maintenir le péage sur le réseau, comme cela a été le cas avant 2006. 2006. Il ne pourrait tout simplement pas faire autrement, les autoroutes n'étant pas amorties à ce jour, sans compter les investissements que nécessiterait l'entretien des services, des infrastructures, des ouvrages et chaussées. Comment assurer alors la sécurité et la pérennité de ce réseau ? Il me semble donc inenvisageable de revenir sur le système des concessions, qui a permis de développer en quelques dizaines d'années dans notre pays un réseau autoroutier dense et moderne, qui est un excellent vecteur touristique. Soyons pragmatiques : l'actuelle situation financière et sociale de la France nous oblige à rechercher le consensus le plus réaliste et le plus satisfaisant pour nos concitoyens, mais également pour l'État, afin qu'il ne se trouve pas dans une position qu'il ne pourrait pas assumer. ce dernier doit contrôler de façon précise le respect par les sociétés concessionnaires d'autoroutes de leurs obligations. L'heure doit donc être à la négociation entre l'État et les concessionnaires. lors de vos récents échanges avec les acteurs de la filière, vous avez appelé leur attention, afin que ces sociétés entendent l'attente forte qui s'exprime en faveur du pouvoir d'achat et formulent des propositions à la hauteur, dans le cadre de leurs politiques tarifaire et commerciale. Je pense qu'une négociation sur des abonnements spécifiques en faveur des usagers réguliers effectuant des trajets domicile-travail, pour lesquels les tarifs de péage représentent une lourde charge mensuelle, pourrait constituer un début de réponse satisfaisant. Pour leur part, les sociétés autoroutières préféreraient troquer une négociation ou un gel des tarifs des péages contre un allongement de leurs concessions, plutôt que de consentir des gestes commerciaux ciblés assez improbables. me semble pouvoir être envisagée, même si l'on sait que les discussions seront âpres et difficiles. Cette voie, passant par la méthode de l'adossement, permettrait, ici ou là, un dialogue renouvelé, notamment avec les métropoles, sans création de péages, puisqu'elle se fonde sur un allongement de la durée des concessions. Allonger d'une courte durée des concessions existantes donnerait la possibilité de financer de l'ordre de 1 milliard d'euros d'investissements. Ne serait-ce pas, madame la ministre, la réponse la plus adaptée, tant pour la question des tarifs que pour celle de l'entretien et de la sécurité de nos autoroutes ?

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous examinons aujourd'hui une proposition de loi visant à nationaliser quatorze sociétés concessionnaires d'autoroutes. Il a déjà été rappelé que la privatisation de sociétés concessionnaires d'autoroutes intervenue en 2006 n'avait pas fait l'unanimité, tant s'en faut ... C'est sans doute ce qui a motivé nos collègues du groupe communiste républicain citoyen et écologiste à rédiger ce texte. Bien sûr, nous sommes d'accord sur le constat : la situation actuelle n'est pas satisfaisante. de façon tout aussi évidente, nous sommes en désaccord sur la temporalité de cette proposition de loi, qui n'est pas opportune. Débourser 50 milliards d'euros pour nationaliser des sociétés- dont certaines verront leur concession expirer dans les vingt prochaines années -nous paraît non seulement déraisonnable, mais aussi irréaliste. Où trouver l'argent ? Ah ! La France doit-elle s'endetter plus encore ?

Le Gouvernement est par ailleurs engagé dans un grand et beau chantier : le fameux projet de loi d'orientation des mobilités, dit LOM. Dans une dizaine de jours, nous aurons un débat en séance publique, qui traitera notamment des autoroutes et des projets d'infrastructures, mais mais pas de leur mode de gestion, ce que nous regrettons. Ce débat est opportun non pas aujourd'hui et pour demain, mais demain pour dans quinze ou vingt ans, lorsque les concessions arriveront progressivement à leur terme. Il faut bien l'admettre la privatisation n'est pas la meilleure idée que nous ayons eue il y a treize ans, non seulement parce que le prix des cessions a largement été sous-estimé selon le rapport établi en 2009 par la Cour des comptes, mais aussi parce que les contrats de concessions se sont révélés extrêmement « piégeants » pour l'État. Cette privatisation fut bien une bonne affaire, mais pas pour l'État ! Au moment même où la très grande partie du réseau est déjà bâtie, la rentabilité de ces infrastructures ne fait qu'augmenter

L'Autorité de la concurrence a indiqué dans son avis de 2014 que les sociétés concessionnaires d'autoroutes affichaient une rentabilité exceptionnelle qui ne se justifiait ni au regard de leurs coûts ni au regard des risques pesant sur elles. Par ailleurs, la réalisation des travaux sur les tronçons concédés a suscité une vive inquiétude, puisqu'ils sont souvent effectués par des entreprises liées aux sociétés concessionnaires. Cette pratique est de nature à augmenter le prix de ces travaux, d'abord, parce que la concurrence s'en trouve réduite, ensuite, parce que le montant des travaux donne lieu à des contreparties de la part de l'État, allant d'une hausse supplémentaire des péages à l'allongement des concessions consenties. Les sociétés concessionnaires pourraient succomber à la tentation d'augmenter les prix des travaux réalisés par des sociétés amies ! À cette situation s'ajoute l'augmentation constante des péages - plus de 20 % depuis la privatisation. Nous en sommes relativement protégés dans les Hauts-de-France,

La plupart des autoroutes sont en effet payantes et les augmentations des tarifs sont très difficiles à endiguer. En 2015, l'État a tenté de geler leur hausse, mais cela a été fait en violation des contrats de concessions. Pour cette raison, à partir de cette année et pour les quatre prochaines années, l'usager paiera, en plus de l'augmentation annuelle classique, une augmentation dont le produit équivaudra à 500 millions d'euros. Nous regrettons d'autant plus vivement le manque de vision stratégique de l'État sur ce dossier- de la privatisation de 2006 au suivi aléatoire des concessions accordées aux sociétés d'autoroutes -que ce manque de vision aboutit à des conséquences malheureuses pour les usagers, les Français. Dans ce contexte, le rôle de l'Arafer doit être renforcé pour plus de transparence et de concurrence et pour réduire ces dommages collatéraux. Le groupe Les Indépendants ne votera donc pas cette proposition

et qui doit évoluer, madame la ministre, pour réduire les conséquences incroyables pour l'État et pour les usagers ; il l'est surtout pour les prochaines années, lorsqu'il s'agira de reposer la question du mode de gestion de ces infrastructures stratégiques. Le débat que nous aurons prochainement sur le projet de loi LOM sera, nous l'espérons, l'occasion de poser les bases de ces réflexions. La parole est à M. Frédéric Marchand.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans moins de deux semaines, nous commencerons l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités. Pourtant, il faut croire que l'impatience de nos collègues du groupe CRCE était trop grande, puisque nous avons à débattre aujourd'hui d'un sujet essentiel s'agissant de mobilités, les autoroutes, même si notre discussion reste très arc-boutée programmée depuis décembre ! Le sujet des autoroutes est extrêmement sérieux, mais, pour démarrer cette intervention, vous me permettrez cette légèreté en citant un humoriste français à la gauloiserie bien connue : « C'est un scandale. J'ai pris l'autoroute à contresens et on ne m'a même pas remboursé. Cette saillie comique illustre bien le débat qui existe aujourd'hui dans notre pays s'agissant des péages acquittés et du retour pour l'État. Concernant les réseaux autoroutiers, vous le savez, l'État a commencé à céder ses parts en 2001, la privatisation s'imposant quant à elle en 2006 face à un bilan alarmant : il s'agissait alors de faire face à 30 milliards d'euros d'endettement. Le Gouvernement déclenchait la privatisation, pour un prix d'achat de 22,5 milliards d'euros. Il faut noter que, en 2009, un rapport de la Cour des comptes affirmait toutefois que ce prix avait été sous-évalué, non non de 10 milliards d'euros comme cela nous est indiqué, mais de 1,5 milliard d'euros au regard d'une valeur estimée à 24 milliards d'euros. Les entreprises qui ont remporté le marché ont connu une forte augmentation de leurs profits, non seulement au travers d'une augmentation des tarifs de péage dont on nous dit qu'elle est de 20 % en dix ans sans que ces chiffres aient été vérifiés, ce qui pose question, mais également grâce à l'automatisation massive des péages, avec pour conséquence l'augmentation du montant des redevances autoroutières. Le financement de l'Afitf, sujet sur lequel nous reviendrons dans le cadre de l'examen du projet de loi LOM, a bien évidemment été touché par cette décision avec près de 15 milliards d'euros depuis sa création en 2005 fléchés en recettes. Le droit des sociétés concessionnaires à percevoir le péage en contrepartie de la construction, de l'extension, de l'entretien et de l'exploitation de leur réseau constitue le fondement du contrat de concession autoroutière. Ce contrat qui lie le concessionnaire et l'État, en particulier le cahier des charges qui lui est annexé, définit le cadre strict d'évolution des tarifs. Ce système contractuel est établi sur la base d'un équilibre financier, prévoyant une évolution annuelle des tarifs de péages jusqu'à la fin de la concession. vifs débats qui ont visé le secteur autoroutier depuis 2013, un accord a été trouvé au mois d'avril 2015 pour rééquilibrer les relations entre les concessionnaires et l'État. Cet accord s'est notamment traduit par un gel des tarifs, mais avec un report de la hausse sur les années 2019 à 2023, le versement par les sociétés d'autoroutes d'un milliard d'euros au au profit de l'amélioration des infrastructures de transport du pays et la réalisation par les sociétés d'autoroutes d'un programme de plus de 3 milliards d'euros de travaux afin d'améliorer le réseau autoroutier en échange d'un allongement de la durée des concessions de deux ans et demi en moyenne, parfois de Cette même année, l'Araf, créée en 2009 pour veiller au bon fonctionnement du marché ferroviaire, a vu ses missions étendues au transport interurbain et aux autoroutes sous concessions, devenant ainsi l'Arafer. de septembre 2016, le ministre chargé des transports annonçait un nouveau plan autoroutier, qui prévoyait un milliard d'euros d'investissements dans les infrastructures autoroutières moyennant une hausse de 0,4 % des péages entre 2018 et 2020. La mesure a été réétudiée par le Gouvernement après un avis sévère de l'Arafer. finalement lancé en 2018 : il s'agit d'un investissement de 700 millions d'euros, financé par une hausse tarifaire comprise entre 0,1 % et 0,4 %, mais aussi par les collectivités locales.

Sans doute faudra-t-il insister sur la nécessaire négociation des tarifs avec les sociétés autoroutières dans le cadre établi. S'agissant de la proposition qui nous est soumise, les estimations du coût de la renationalisation immédiate des sociétés d'autoroutes

D'ailleurs, dans le contexte du mouvement des « gilets jaunes », qui est né des contestations du coût élevé des transports, la ministre des transports a appelé les concessionnaires à des gestes commerciaux. Cependant, il s'agit d'un appel à la bonne volonté. Rien de contraignant n'a été mis en place pour le moment, mais c'est sans doute une piste qu'il ne faut pas s'interdire de creuser.

En revanche, il nous faut avoir à l'esprit l'échéance de 2033 et imaginer d'ores et déjà les scénarios et solutions pour trouver les réponses les plus pertinentes pour l'État, pour nos concitoyens, sans oublier bien évidemment les sociétés autoroutières. Pour toutes ces raisons, vous comprendrez que le groupe La République En Marche votera contre ce texte.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, voilà quelques semaines, une large majorité s'est dégagée ici, indépendamment des clivages politiques, pour s'opposer à la privatisation d'Aéroports de Paris. Ce vote a été largement salué dans le pays. L'exemple de la privatisation des autoroutes était alors dans toutes les têtes et son échec sur toutes les lèvres. Je me souviens que, du côté droit de l'hémicycle, on a même fort justement affirmé que cette privatisation avait été une expérience « catastrophique En cohérence, notre groupe a souhaité remettre le sujet de la nationalisation des autoroutes au coeur de nos discussions. La proposition de loi que nous proposons mérite d'être examinée sans idéologique. Elle invite d'abord à s'interroger sur le rôle de l'État dans l'aménagement du territoire. L'État n'est aujourd'hui plus en mesure de faire prévaloir l'intérêt général face à la puissance des sociétés concessionnaires le droit des contrats passés devient plus fort que la souveraineté politique. Dernier exemple en date, à mes yeux parmi les plus choquants, l'exonération de péages votée pour les véhicules de secours devrait, selon ces contrats, conduire à une indemnisation par l'État des sociétés concessionnaires. Pour cette raison, cette exonération ne sera pas appliquée et les véhicules de police, des pompiers ou du SAMU continueront de s'acquitter des péages

L'État a organisé sa propre incapacité à mettre en place une tarification sociale ou environnementale, à oeuvrer en faveur de la complémentarité entre modes de transport et à réaliser le report modal du routier vers le ferroviaire. La privatisation est aussi une aberration économique aux conséquences lourdes. On peut débattre à l'infini des chiffres des bénéfices et des dividendes perçus et distribués par les sociétés concessionnaires. Il reste qu'il y a bien un consensus

Les autoroutes sont donc un bien économiquement viable permettant, sans prise de risques, d'obtenir d'importants bénéfices. Or cet argent ne tombe pas de nulle part. C'est celui des Français, qui subissent la hausse des tarifs, laquelle, après une accalmie, a repris au mois L'État lui aussi continue d'être mis à contribution, tout comme les collectivités territoriales. Ces dernières participent notamment aux investissements lorsqu'il s'agit de construire de nouvelles bretelles raccordant les territoires au réseau autoroutier. J'en connais des exemples en Normandie, mais chacun d'entre nous pourrait en citer Nationaliser les autoroutes permettrait donc d'utiliser ces bénéfices pour l'intérêt général en permettant à l'État de trouver de nouvelles ressources pour le financement des infrastructures. L'Agence de financement des infrastructures de transport de France a en effet été privée de ressources pérennes par la privatisation, ce qui l'empêche d'assumer son rôle, aussi bien pour favoriser la mobilité sur tout le territoire que pour permettre le report modal nécessaire à l'urgence écologique et à la sécurité routière. Alors que nous nous apprêtons à débattre dans les prochains jours du projet de loi d'orientation des mobilités, dont la programmation est totalement sous-financée, il serait judicieux de s'appuyer sur une source pérenne de financement plutôt que sur un doublement des recettes des radars, comme l'ont évoqué certains de nos collègues. Enfin, et peut-être surtout, il est nécessaire d'assumer le caractère politique de cette question. Les « gilets jaunes », à la suite de nombreuses associations d'usagers qui agissent en ce sens depuis des années, se sont chargés de nous le rappeler. La nationalisation des autoroutes fait partie de leurs principales revendications, comme en témoignent les nombreuses opérations « péage gratuit ». Ce que les « gilets jaunes » ont aussi rappelé, c'est que l'organisation actuelle du système autoroutier ne fonctionnait pas : entre ceux qui ne peuvent se permettre d'emprunter les autoroutes trop chères, ceux pour qui ces dépenses ne cessent de peser dans le budget et ceux qui sont tout simplement exclus du réseau autoroutier, les Français ont tordu le cou à cette conception technocratique et coupée des réalités sociales selon laquelle tout va bien tant que les autoroutes sont bien entretenues. Je précise d'ailleurs que la comparaison entre l'état des autoroutes et celui des routes secondaires plaide, elle aussi, pour la nationalisation. En effet, si les sociétés gestionnaires ont les moyens de réaliser les travaux nécessaires, c'est bien parce qu'elles bénéficient d'une source de financement que n'ont pas les routes secondaires. La nationalisation permettrait donc une redistribution plus favorable au réseau secondaire. Les revendications de la population sont très claires : on ne veut pas d'une renationalisation dans dix, vingt ou trente ans, au risque très probable que les contrats actuels soient reconduits jusqu'à constituer une privatisation indéfinie de fait. Non ! On veut simplement arrêter de payer dès maintenant pour un service qui devrait être public et qui sert des intérêts particuliers. Mes chers collègues, montrez à nos concitoyens que vous n'êtes pas sourds à leurs revendications et que vous souhaitez répondre au vent de colère qui souffle dans notre pays. Avec nous, votez la nationalisation des autoroutes ! La parole

C'est un sujet qui suscite- à juste titre -de nombreuses interrogations, voire de la défiance chez nos concitoyens. Le groupe Union Centriste avait proposé un débat parlementaire sur ce sujet qui, malheureusement, a dû être reporté en raison de la manifestation contre l'antisémitisme. Voilà maintenant plus de douze ans, l'État privatisait ses autoroutes pour des concessions de trente ans en moyenne. On nous indiquait à l'époque qu'il s'agissait d'une « bonne affaire » pour l'État, donc pour le contribuable. L'ensemble des privatisations rapportait 14,8 milliards d'euros. Or, en douze ans, les sociétés d'autoroutes ont déjà versé à leurs actionnaires 14,9 milliards d'euros. En 2017, l'ensemble de ces sociétés ont dégagé 73 % de marge brute ! Je serais curieux de savoir s'il existe, en France, une entreprise qui peut en faire autant. La renationalisation proposée aujourd'hui est estimée à 50 milliards d'euros, vous l'avez souligné, madame la ministre, soit le triple de ce qu'ont rapporté les privatisations ... Une bonne affaire pour le contribuable ? Certainement pas ! Où est également la bonne affaire pour les usagers de l'autoroute ? Selon les chiffres à notre disposition, dont on ne peut pas dire qu'ils soient marqués du sceau de la transparence, le chiffre d'affaires de ces sociétés augmente beaucoup plus vite que le trafic. Son augmentation découle donc essentiellement de l'augmentation du tarif des péages. Les usagers ont vu les prix des péages s'envoler ; les augmentations ont été plus fortes que l'inflation. L'usager a donc perdu du pouvoir d'achat. En plus, l'évolution des tarifs des péages ne semble pas prise en compte dans l'indice de l'Insee de calcul de l'inflation. les automobilistes dépensent désormais autant en péage qu'en carburant sur un nombre de plus en plus grand de trajets. Pourtant, si le service fourni est bon, il ne s'est pas nettement amélioré. Ce qui est certain, c'est que l'on n'a jamais construit aussi peu d'autoroutes que depuis la privatisation. Entre 2007 et 2013, seulement 167 nouveaux kilomètres ont été réalisés, alors que le réseau kilomètres. Comme s'il n'était pas suffisant de vendre la poule aux oeufs d'or et de l'alimenter au détriment de l'usager, on organise ce jeu de dupe dans le dos des Français. Je veux parler ici de l'accord secret conclu en 2015 entre Mme Royal et les sociétés d'autoroutes. En contrepartie d'un pseudo-gel des tarifs pour 2015, les sociétés autoroutières ont obtenu de nouvelles hausses tarifaires jusqu'en 2032, l'engagement de l'État de compenser toute modification fiscale ou obligation nouvelle, la prolongation des concessions de deux à cinq ans.

En tout cas, l'accord de 2015 est toujours officiellement secret, en attendant que le Conseil d'État ne se prononce sur le bien-fondé de sa confidentialité. Pourquoi un tel secret ? Était-ce pour cacher aux Français que, en matière d'autoroutes, leurs intérêts étaient, une fois de plus, sacrifiés au profit de ceux des sociétés d'autoroutes ? Malgré les lourdes critiques que je viens d'énoncer, une renationalisation anticipée des autoroutes me semble juridiquement dangereuse et très lourde financièrement. Il est d'ailleurs complètement incohérent de faire supporter ce coût aux entreprises un relèvement de l'impôt sur les sociétés : c'est là un contresens économique. En outre, nous ne sommes pas certains que l'État serait en capacité d'assurer un entretien des autoroutes équivalent à ce qui se fait aujourd'hui. N'oublions pas que les autoroutes sont l'une des vitrines de la France et que l'État ne se révèle pas souvent bon gestionnaire. Nous continuerons toutefois de demander au Gouvernement de faire la lumière sur les relations entre l'État et les sociétés autoroutières. Il est temps d'arrêter les accords secrets contre des allongements injustifiés de concession. La parole

Les vicissitudes de la vie parlementaire que nous connaissons avec plus ou moins d'acuité nous amènent trop souvent à examiner des dispositions non normatives ou qui ne relèvent pas du domaine de la loi. Dans d'autres cas, le Gouvernement, comme il le fait désormais à chacun de ses grands textes, nous enjoint de consacrer dans la loi des objectifs dont nous savons qu'ils ne seront jamais atteints. Puis, il y a toutes ces fois où nous sommes contraints de voter des dispositions parce que tel décret d'application ou telle interprétation jurisprudentielle nous y aura conduits. Difficile dans ces conditions d'être trop ambitieux et difficile, surtout, de faire de la politique. Avec cette proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes et à l'affectation des dividendes à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France,

S'agissant de l'exposé des motifs, je peux m'associer à nombre de postulats qui y sont formulés. Je souscris à l'insécurité engendrée par les privatisations sur les ressources de l'Afitf. Je souscris à l'analyse qui est faite sur l'utilisation du produit de la vente, produit qui a été utilisé en vue du désendettement de l'État. Je souscris à l'analyse relative au gel des tarifs décidé en 2015. Je souscris enfin à l'analyse sur la rentabilité financière des sociétés concessionnaires, analyse adossée au rapport de la Cour des comptes de 2013 et à l'avis de l'Autorité de la concurrence de 2014. Je rappelle au passage que ces deux institutions n'ont pas exactement la même appréciation. appréciation. Je ne compte pas entrer dans le débat sur le rachat des contrats de concession, car telle est la question en dernier ressort de ce texte. Encore une fois, je comprends la démarche intellectuelle qui consiste à dire que l'exercice politique ne doit pas systématiquement conduire à l'impuissance publique, mais je ne veux pas entrer dans un débat sur l'évaluation économique d'une opération de rachat que les auteurs de la proposition de loi et que plusieurs d'entre nous évaluent entre 28 et 50 milliards d'euros et que le Sénat évaluait, pour sa part, entre 30 et 40 milliards

qui était membre du groupe CRCE. À l'époque déjà, nos analyses étaient convergentes. Je ne souhaite pas non plus alimenter un débat sur l'état de la jurisprudence en matière de libéralités. Compte tenu de l'ampleur de l'opération, nous avancerions en plein brouillard.

lors de la table ronde sur l'état des infrastructures routières et autoroutières du 8 février 2017, organisée par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, lors des conclusions du groupe de travail de notre commission sur les sociétés concessionnaires d'autoroutes le 17 décembre 2014, et même lors de l'examen de la proposition de loi relative à la nationalisation des sociétés concessionnaires d'autoroutes et à l'affectation des dividendes

mais une fois que ces concessions seront arrivées à échéance, dans les années 2030, nous voulons que l'État puisse étudier l'ensemble des possibilités qui s'offriront alors conserver un régime concessionnaire en introduisant des garanties, comme celles qu'a proposées le groupe de travail précité, en mettant fin à la pratique des contrats de plan, en abaissant le seuil de mise en concurrence des marchés de passation de travaux ou en élargissant les compétences de l'Arafer

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans un rapport de juillet 2013 portant sur les relations entre l'État et les sociétés concessionnaires d'autoroutes, la Cour des comptes consacrait un chapitre entier à l'insuffisante régulation des hausses de tarifs. Elle relevait notamment que le décret de 1995 relatif aux péages autoroutiers ne garantissait pas une protection suffisante des intérêts du concédant et des usagers. Elle jugeait par ailleurs que l'État avait accordé aux concessionnaires de compenser par des hausses de tarifs un grand nombre d'investissements de faible ampleur, dont l'utilité pour l'usager n'était pas toujours avérée, ou qui relevaient de leurs obligations normales. Dans un avis du 17 septembre 2014, après avoir constaté que le chiffre d'affaires des sociétés concessionnaires d'autoroutes avait augmenté beaucoup plus fortement que la progression du trafic, l'Autorité de la concurrence formulait plusieurs préconisations pour une meilleure régulation du secteur, portant notamment sur les modalités de fixation des tarifs des péages et sur une amélioration des conditions de la concurrence dans les appels d'offres pour les travaux de rénovation et d'extension du réseau. Les articles 5 et 6 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont venus renforcer les prérogatives de l'Arafer sur l'ensemble de ces sujets. En effet, un mécanisme correcteur en cas de bénéfices supérieurs aux estimations a été introduit. La transparence a été améliorée avec la publication des contrats entre l'État et les sociétés d'autoroutes. L'Arafer a publié en juillet 2018 son rapport annuel sur les marchés et les contrats passés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en 2017, soit la première année de pleine d'application du nouveau cadre régulatoire. Elle constate que « la majorité des achats- en montant -des sociétés concessionnaires fait aujourd'hui l'objet d'une procédure transparente et objective de mise en concurrence au bénéfice de l'ensemble des opérateurs économiques Dans son rapport annuel de novembre 2018 sur la synthèse des comptes des concessions autoroutières, l'Arafer relève à propos des hausses tarifaires que : « L'effet des hausses spécifiques- liées à la compensation de la redevance domaniale ou à la compensation d'investissements supplémentaires prévus par les contrats de plan -s'est atténué sur la période. Les hausses tarifaires restent toutefois plus dynamiques que l'inflation de référence. » Ce rappel historique illustre à quel point il est important de prévoir un cadre régulatoire précis et contraignant concomitamment à la décision de privatiser des actifs publics, d'autant plus lorsqu'ils sont en situation de monopole. Alors que l'Assemblée nationale débat en seconde lecture du projet de loi Pacte, je ne peux manquer d'attirer l'attention des députés sur le renforcement de la régulation du secteur aérien prévu aux articles 47 et 48, tels qu'ils ont été votés par le Sénat sur l'initiative du rapporteur Jean-François Husson. Si les dispositions de l'article 48 issues des travaux de l'Assemblée nationale ont quelque peu renforcé les pouvoirs de l'État à l'occasion de la renégociation de ces contrats ou en leur absence, ceux-ci demeurent insuffisants pour faire prévaloir l'intérêt général en cas de conflit avec le futur propriétaire privé d'Aéroports de Paris. C'est pourquoi le Sénat a prévu de donner la possibilité à l'État d'adopter unilatéralement un quasi-contrat de régulation économique en cas de désaccord persistant avec ADP ou encore d'imposer à ADP la réalisation d'investissements nécessaires au respect des obligations de service public. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, à l'instar de mon groupe, je voterai contre cette proposition de loi visant à renationaliser les autoroutes. Laissons le temps Laissons le temps faire son oeuvre avant de vouloir de nouveau rebattre les cartes : le nouveau cadre régulatoire est encore bien récent. Ayons en tête cette expérience, au moment où il est envisagé de privatiser d'autres infrastructures de transport.

la mise en oeuvre de la clause sur les surprofits qui a été introduite dans le cadre du plan de relance autoroutier. L'évaluation de la rentabilité des sociétés d'autoroutes sera

de 10,14 %. Les séquences tarifaires prévues dans les contrats de concession sont de 70 % de l'inflation ou de 85 % de l'inflation lorsqu'il existe un contrat de plan prévoyant par ailleurs des investissements à la charge de la société concessionnaire.

je tiens à remercier nos collègues, quelques jours après le débat sur Aéroports de Paris, qui avait donné lieu ici à un beau rassemblement transpartisan,

ce sont de nombreuses rentrées d'argent pour le ministère des finances : la taxe autoroutière, la récupération de la TVA et l'impôt sur les sociétés. Bref, c'est une vache à lait à

Qui peut penser que nous maîtriserons nos politiques de mobilité, à l'heure de la nécessaire transition écologique, en continuant à écarter de la maîtrise publique des infrastructures aussi majeures ?

nos concitoyens, comme en témoignent les actions qui ont été menées au cours de ces dernières semaines sur les autoroutes, et ce alors que les tarifs des péages ont encore augmenté. L'existence d'une rente autoroutière est aujourd'hui un fait avéré. un fait avéré. Un fort décalage existe entre les tarifs appliqués et les coûts engendrés par le fonctionnement et l'exploitation des autoroutes. Compte tenu du faible niveau de risque lié à l'activité et des besoins en investissements, cette rentabilité n'a pas de justification économique ou sociale.

l'État ne s'étant pas donné les moyens, humains notamment, d'exercer une régulation efficace des concessions autoroutières. De plus, on ne saurait occulter la responsabilité des gouvernements ayant négocié cette privatisation à des conditions particulièrement défavorables. La Cour des comptes l'a rappelé en 2008

elle avait calculé une rentabilité à l'instant des concessions autoroutières en occultant le prix de rachat et la reprise de la dette. Bien évidemment, cela a fait un scandale,

Quand bien même il faudrait investir, la puissance publique peut s'en donner les moyens, d'autant que ce sont les péages qui financeront le remboursement de cet emprunt. Mes chers collègues,

un réseau autoroutier me paraît beaucoup plus proche de l'intérêt public, et, au demeurant, rentable. Je le reconnais, les signatures des contrats de concession ont été tellement favorables aux entreprises que la nationalisation est techniquement

quotidien. Ainsi, les attentes sont fortes pour la réalisation de voiries de contournement adaptées aux évolutions démographiques de nos agglomérations.

2,1 euros au remboursement de la dette et à la rémunération des investisseurs et, enfin, 2,5 euros à la construction et à la modernisation du réseau. Si la gestion des autoroutes était nationalisée, comme le souhaitent les auteurs de ce texte, le quart des recettes des péages affecté à la construction et à la modernisation tomberait dans le tonneau des Danaïdes de Bercy, au détriment de l'entretien et de l'investissement.

Il est donc proposé de supprimer cet article, car la concession reste le seul moyen pour que notre réseau autoroutier demeure un modèle de sécurité, de qualité et de confort reconnu dans toute l'Europe.

que nous opposent nos collègues pour justifier le vote de cet amendement. Éliane Assassi l'a fort bien démontré, c'est une question de choix politique

Le scrutin est ouvert.

tard. Dans la discussion générale, la parole est à Mme Éliane Assassi, auteure de la proposition de loi.

et à proposer une nouvelle doctrine de maintien de l'ordre intervient à un moment critique de la vie démocratique de notre pays, théâtre d'un mouvement citoyen et social d'une longévité sans précédent et d'un caractère totalement inédit. Le mouvement des « gilets jaunes », toujours soutenu sur le plan des revendications par une nette majorité de nos concitoyennes et concitoyens, n'a pas reçu de réponse de long terme à des exigences que nous considérons comme légitimes.

politique. Elle ne saurait être une réponse d'autorité, d'utilisation de la force. En un mot, la répression ne pourra calmer la colère ni l'exaspération ; tout montre au contraire qu'elle ne peut que les attiser. Or, monsieur le secrétaire d'État, après le constat d'une répression accrue des mouvements sociaux ces dernières années, notamment à l'occasion du mouvement contre la loi El Khomri, nous assistons depuis novembre à une tentative d'utiliser la force brute, symbolisée par les LBD 40, pour canaliser ou éteindre un mouvement populaire. Avant d'entrer dans le détail de notre argumentation, je souhaite affirmer fortement notre attachement à une police républicaine, à des forces de l'ordre qui mettent tout en oeuvre pour assurer la sécurité des biens et des personnes. Nos forces de l'ordre sont prises au piège de l'entêtement à maintenir une politique profondément impopulaire et rejetée massivement. La stratégie de la tension, du pourrissement, n'est pas la bonne. elle n'a pas toujours été celle choisie par les autorités policières : comment ne pas rappeler l'attitude responsable et courageuse du préfet Grimaud, qui, en 1968, n'a pas jeté de l'huile sur le feu et a préservé au maximum Paris d'affrontements sanglants et mortels ? Il ne s'agit pas pour nous de mettre en cause collectivement les fonctionnaires de police, qui, la plupart du temps et majoritairement, sont piégés entre les exigences insatisfaites des manifestants et les ordres venus d'en haut- de vous, monsieur le secrétaire d'État -, le tout dans un climat d'épuisement. C'est dans ce cadre que, depuis le 17 novembre, le volume de tir des armes dites intermédiaires atteint un niveau critique. Critique est également le nombre de personnes blessées, souvent gravement, à la suite de l'utilisation de ces armes.

armes à feu et armes de guerre. C'est une arme non létale si elle est utilisée dans les conditions préconisées par le constructeur, conditions qui ne sont pas toujours appliquées.

L'utilisation des lanceurs de balles de défense doit nous poser question. Au-delà des atermoiements de l'exécutif, nous nous interrogeons sur le nombre de victimes qu'il faudra encore avant qu'on légifère sur l'usage de cette arme. Nous refusons la banalisation actuelle de blessures très graves, des blessures qui atteignent la République de plein fouet. Notre pays peut-il accepter encore ces scènes sanglantes ? Au cours de nos auditions et tables rondes, nous avons constaté qu'aucune arme ne peut réellement sécuriser les manifestations et ceux qui les encadrent. Il convient, dès lors, de réfléchir à la globalité du dispositif. C'est ainsi que nous proposons un triptyque de mesures. D'abord, nous demandons l'arrêt immédiat de l'usage des lanceurs de balles de défense, pour cause de santé publique et d'atteintes graves à l'intégrité physique des manifestants. voulons une plus grande transparence des données relatives à l'usage des armes. Sans le travail des journalistes et spécialistes sur la question, nous n'aurions aucun chiffre fiable- l'exécutif ayant attendu des semaines -sur l'utilisation de ces armes. Or le manque de transparence du pouvoir nuit autant à notre démocratie qu'à l'analyse de la situation. Enfin, il est temps de mener une réflexion poussée sur nos doctrines de maintien de l'ordre et de formation des forces de sécurité. Nous souhaitons que s'engage à cet égard une réflexion à long terme : nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport détaillé et documenté sur les stratégies de désescalade et de pacification à mettre en oeuvre dans le cadre du maintien de l'ordre. Nous pouvons nous appuyer sur de nombreux exemples européens pour revoir notre doctrine

aux conditions de travail des agents, qui ne sont pas assez formés et se retrouvent démunis face à un climat de tension qui ne cesse de s'intensifier. Ainsi, l'usage exagéré des lanceurs de balles de défense produit l'effet inverse de sa vocation : il représente le premier obstacle entre forces de l'ordre et manifestants. Aujourd'hui, il faut donc dire « stop » au LBD 40. C'est une mesure d'urgence ! En effet, même si la doctrine d'emploi de cette arme et son encadrement juridique sont précis,

d'absolue nécessité, n'est vérifié en pratique ni par les manifestants ni par les journalistes présents. Les ordres donnés, la désorganisation et le manque de formations sont, pour une bonne part, à la source des difficultés. Les effectifs de policiers et gendarmes formés aux situations de maintien de l'ordre ne sont pas suffisants. Résultat : on doit recourir à l'emploi d'unités dont ce n'est pas la fonction. Je pense notamment aux unités formées à la lutte contre les violences urbaines, les brigades anti-criminalité : elles sont formées à l'interpellation, non à l'action collective pour circonscrire les débordements de manifestants. Sur les 13 460 tirs de balles de défense effectués par toutes les unités de la police nationale, 85 % sont dus aux unités civiles présentes sur le périmètre, non aux CRS, dont le maintien de l'ordre et l'utilisation des LBD 40 dans ce cadre sont la fonction. Pis, de l'aveu de certains policiers, des LBD sont mis entre les mains d'agents qui n'ont jamais touché une arme, notamment celle-là ... La formation dont nous parlons, hors unités spécifiques de maintien de l'ordre, consiste à tirer cinq balles tous les trois ans, sans mise en situation réelle ni cible mouvante. Nos manifestations sont donc encadrées par des agents qui ne sont pas formés au maintien de l'ordre et dont on peut douter qu'ils maîtrisent l'arme qu'ils portent. Les unités sont disparates et épuisées ; leur commandement entre compagnies n'est pas unifié, et elles se gênent mutuellement. Des policiers nous ont dit On nous fait faire des erreurs », « la BAC nous gêne dans notre action », « sur le terrain, nous n'avons aucune vision d'ensemble », « nous n'avons pas l'impression de commettre des actes illégaux ». Le manque d'effectifs et de formation des forces de l'ordre perturbe gravement la stratégie traditionnelle d'évitement entre la police et les manifestants. un seul bilan : la mise en danger des forces de l'ordre et des manifestants. Ces conditions de travail inadmissibles pèsent sur nos forces de l'ordre et créent des drames dans nos rues. Nous avons été alertés de nombreuses fois sur l'usage des lanceurs de balles de défense, dès 2009, une pétition en ligne. Sur le terrain législatif, une proposition de loi, déposée la année, visait l'interdiction des armes de quatrième catégorie, dont le flash-ball, contre les attroupements et les manifestations. Nous avons mis en débat, en 2015, notre proposition de loi visant à instaurer un moratoire sur l'utilisation et la commercialisation d'armes de quatrième catégorie et à interdire leur utilisation par la police et la gendarmerie contre les attroupements ou manifestations. Nombreux sont celles et ceux qui se mobilisent pour dénoncer les conditions d'usage et les répercussions du LBD 40. Après plusieurs rapports de la CNDS, le Défenseur des droits recommande d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense

Le 14 février, des experts de l'ONU ont dénoncé l'usage excessif de la force lors des manifestations. Le Conseil de l'Europe et sa commissaire aux droits de l'homme ont suivi. Hier, c'est Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations unies, qui a exigé une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force.

le Sénat est conduit à se prononcer sur un sujet qui, depuis quelques semaines, divise dans le débat public : l'usage des lanceurs de balles de défense dans les opérations de maintien de l'ordre. Notre débat s'inscrit dans un contexte de fortes tensions, que nous ne saurions ignorer dans le cadre de nos échanges. En effet, voilà maintenant seize semaines que nous assistons, sur l'ensemble du territoire, à des manifestations hebdomadaires qui s'accompagnent d'actes de violence et de dégradations sans précédent. Outre des dégâts matériels d'une ampleur inédite, un nombre malheureusement important de blessés est à déplorer, du côté des manifestants comme des forces de l'ordre. Dans ce contexte pour le moins inédit, beaucoup s'interrogent, légitimement, sur l'adéquation de la doctrine française de maintien de l'ordre. Il est certain que les événements récents appelleront des évolutions. C'est d'ailleurs dans cette optique que le Sénat a adopté, dès le mois d'octobre dernier, une proposition de loi visant à prévenir et sanctionner les violences lors des manifestations, proposition qui reviendra en discussion dans notre hémicycle La proposition de loi soumise à notre examen s'inscrit assurément dans ce débat, mais elle adopte un angle précis, en mettant l'accent uniquement sur la réduction de l'usage de la force par les forces de l'ordre.

loi vise ensuite à renforcer la transparence sur l'usage des armes par les forces de l'ordre, en ouvrant au public le traitement relatif à l'usage des armes, qui recense l'ensemble des cas d'usage par les agents de police. Enfin, elle prévoit la remise d'un rapport au Parlement sur les avantages et les inconvénients de chaque type de doctrine au niveau européen et sur les alternatives à mettre en oeuvre dans notre pays pour pacifier le maintien de l'ordre dans le cadre des manifestations. S'il soulève un débat essentiel, ce texte n'en présente pas moins d'importantes limites, qui ont conduit la commission des lois à ne pas l'adopter. Avant même de se pencher sur l'opportunité des dispositifs proposés, notre commission a relevé que le texte soulevait des difficultés d'ordre juridique. En effet, la plupart de ses dispositions ne relèvent pas du domaine de la loi, mais du domaine réglementaire. Ainsi en est-il de la liste des armes susceptibles d'être utilisées dans le cadre du maintien de l'ordre, ainsi que des conditions d'accès au fichier relatif à l'usage des armes. Surtout, il est apparu à notre commission que les dispositifs proposés présentaient des difficultés importantes sur le fond. Avant tout, il me semble nécessaire de s'attarder quelques instants sur le cadre juridique d'usage du LBD, qui fait trop souvent l'objet d'approximations. Le LBD ne constitue pas, contrairement aux idées reçues, une arme en libre-service, utilisée à la légère. Bien au contraire, comme l'a rappelé récemment le Conseil d'État, son emploi dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre est strictement encadré. ... De fait, deux usages précis sont prévus par le code de la sécurité intérieure. Le premier, dit collectif, est spécifique aux opérations de maintien de l'ordre : le recours au LBD est autorisé lorsque, à l'occasion d'un attroupement sur la voie publique, des voies de fait ou des violences sont commises à l'encontre des forces de l'ordre, ou lorsque celles-ci ne sont pas en mesure de protéger le terrain qu'elles occupent. Le LBD est alors utilisé en groupe, par l'ensemble de l'unité, sur décision du commandement. Le second usage, dit individuel, repose sur le régime général d'usage des armes par les forces de sécurité intérieure : le LBD peut alors être utilisé, y compris dans le cadre d'une manifestation, lorsque l'usage de l'arme létale est légitime. Il s'agit, par exemple, des cas de légitime défense, d'état de nécessité et de périple meurtrier. En revanche, le LBD ne peut pas être utilisé- j'y insiste -par les unités de maintien de l'ordre en vue de disperser un attroupement après sommations. Son usage est purement défensif. Outre ce cadre légal et réglementaire, une instruction fixe de manière claire et précise la doctrine d'emploi du LBD. Elle prohibe notamment le tir à la tête, ainsi que le tir contre des personnes présentant des signes de vulnérabilité. On ne peut nier que l'usage du LBD, jusque-là assez réduit, a beaucoup progressé au cours des dernières semaines, entraînant parfois des blessures importantes. Selon les informations communiquées à la commission, alors que 6 284 tirs de LBD ont été recensés au sein de la police nationale en 2017, 13 460 tirs ont été dénombrés entre le 17 novembre 2018 et le 5 février 2019. Depuis le début des manifestations des « gilets jaunes », un millier de tirs de LBD ont été effectués par les escadrons de gendarmerie mobile, contre une cinquantaine seulement en 2017.

de ne pas confondre l'usage légitime et légal d'une arme, qui est toujours susceptible de blesser, avec le mésusage de la force. Constater des blessures, aussi graves soient-elles, ne suffit pas à établir que l'emploi de l'arme était illégitime. L'existence d'éventuelles dérives personnelles dans l'usage des LBD, qu'il appartient à la justice de condamner fermement, ne justifie pas davantage d'interdire l'emploi l'on ne peut que regretter que l'usage du LBD puisse, dans certaines circonstances, provoquer des blessures parfois d'une gravité certaine, force est de constater que le nombre de blessures liées à des lanceurs de balles de défense demeure réduit par rapport au nombre de tirs effectués. Sur les 13 460 munitions utilisées dans le cadre des manifestations sur la voie publique entre novembre 2018 et février 2019, l'Inspection générale de la police nationale n'aurait été saisie que de cinquante-six cas de graves blessures.

Le lanceur de balles de défense est une arme de force intermédiaire nécessaire à la mise en oeuvre d'une réponse graduée et d'un usage proportionné de la force. En interdire l'usage reviendrait à supprimer un échelon dans l'arsenal des moyens à la disposition de nos forces de l'ordre, avec deux risques : inciter au contact direct entre manifestants et forces de l'ordre, qui n'est pas de nature à réduire le nombre de blessés, et induire un recours plus fréquent à l'arme létale. raisons, la Cour européenne des droits de l'homme exige la mise en oeuvre d'une réponse graduée et d'un usage proportionné de la force dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. Dans un arrêt de 1998, elle a ainsi condamné la Turquie pour n'avoir pas doté ses forces de police d'autres armes que les armes à feu et, ainsi, ne pas leur avoir laissé d'autre choix que d'utiliser leurs armes létales à l'occasion d'une manifestation. Si ces arguments plaident pour le maintien de l'usage du LBD, il demeure toutefois essentiel de s'assurer de la bonne utilisation de celui-ci et du strict respect du cadre juridique. À cet égard, je tire de mes auditions le constat de quelques marges d'amélioration possibles pour perfectionner l'usage du LBD. Tout d'abord, nombreux sont ceux qui appellent à une amélioration de la formation à l'usage de cette arme : l'obligation d'entraînement tous les trois ans est jugée insuffisante par de nombreux policiers et gendarmes. Par ailleurs, si la mise en place de caméras mobiles pour documenter l'usage de cette arme constitue une avancée importante, il m'a été indiqué que des améliorations techniques mériteraient d'y être apportées pour les rendre complètement opérationnelles. Monsieur le secrétaire d'État, ces éléments nous paraissent essentiels : nous sommes intéressés de vous entendre sur les réflexions envisagées par vos services sur le sujet. Pour finir, je résumerai en quelques mots la position de notre commission sur les deux autres articles du texte. texte. Comme l'interdiction du LBD, l'ouverture au public du traitement relatif à l'usage des armes est porteuse de risques pour les forces de l'ordre. Outre les difficultés qu'elle soulève en termes de protection des données personnelles, elle pourrait conduire à rendre publiques des données relatives aux conditions d'intervention des forces de l'ordre, ce qui risquerait de fragiliser leur action. De plus, ouvrir ce traitement ne donnerait qu'une vision partielle de l'usage des armes, car il ne concerne que la police nationale. Enfin, par le biais d'une demande de rapport au Parlement, les auteurs de la proposition de loi invitent à repenser la doctrine française du maintien de l'ordre, en s'inspirant des modèles mis en oeuvre dans d'autres pays européens. Le débat mérite d'être posé. Toutefois, les pistes esquissées par la proposition de loi ne paraissent pas de nature à répondre aux défis auxquels le dispositif français de maintien de l'ordre est aujourd'hui confronté. Contrairement à la conception communément admise, les doctrines fondées sur le principe de désescalade ne sont pas, en pratique, exemptes de tensions avec les forces de l'ordre. Un rapport de 2014 des inspections générales de la police et de la gendarmerie nationales révèle ainsi que la doctrine allemande, souvent citée en exemple, est en réalité fondée sur une entrée en contact rapide avec les manifestants et s'accompagne d'un nombre élevé de blessés.

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, depuis quelques semaines, le débat sur le maintien de l'ordre public se concentre sur une arme non létale employée par nos policiers et gendarmes : le lanceur de balles de défense, plus communément appelé le LBD. Depuis des semaines, l'ordre public connaît des troubles majeurs. Ces troubles illustrent l'évolution à l'oeuvre dans les manifestations de voie publique. De plus en plus, la violence s'infiltre dans les manifestations, qui sont un mode d'expression démocratique, légitime De plus en plus, à côté des manifestants pacifiques, les forces de l'ordre voient surgir des groupes ultraviolents, dont le seul objectif est de casser et de violenter. Matériel urbain, vitrines de magasins, symboles de la République, bâtiments

loi. Je pourrais également citer des événements plus récents, qui ont trait au mouvement dit des « gilets jaunes » : ces motards de la préfecture de police de Paris pris à partie sur les Champs-Élysées, le 22 décembre dernier, ou la scène ahurissante qui s'est déroulée sur la passerelle Senghor, début janvier. Depuis le 17 novembre, il y a eu près de 1 500 blessés parmi les forces de l'ordre, qu'il s'agisse de policiers, de gendarmes ou même de pompiers. Depuis le 17 novembre, on a compté près de 80 dégradations majeures sur des bâtiments publics. Nous ne parlons pas de manifestations pacifiques, déclarées, de gens qui expriment des revendications. Sur le terrain, nous sommes confrontés, policiers, gendarmes, à des individus extrêmement violents qui veulent en découdre et dont c'est apparemment la seule motivation. Ces violences, qui sont inqualifiables,

aux techniques de dispersion classique des cortèges, il faut substituer des techniques destinées à lutter contre des violences urbaines, contre des émeutes. C'est dans ce contexte très particulier que doit se poser la question de l'armement mis à disposition des forces de l'ordre. Or la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui, si elle était adoptée, priverait ces forces de l'ordre d'un moyen devenu nécessaire pour dissiper les violences et contenir les débordements.

Les forces de l'ordre agissent, en effet, dans un cadre légal précis et sont guidées par deux principes fondamentaux : l'absolue nécessité et la stricte proportionnalité, qu'elles interviennent en légitime défense ou pour disperser un attroupement. Il s'agit toujours de contenir les individus les plus agressifs et de les disperser, en évitant d'attiser la violence et en préservant ainsi ceux qui veulent, eux, porter leurs revendications pacifiquement. Jamais ce gouvernement n'a dissuadé de manifester ! La preuve, tous les samedis, nous encadrons des manifestations et des mouvements. anticasseurs ? L'utilisation du lanceur de balles de défense constitue une réponse graduée et proportionnée à la multiplication des situations de danger. Ainsi, lors d'opérations de maintien de l'ordre, il ne peut être fait usage du LBD que si des voies de fait ou des violences sont commises contre les forces de l'ordre ou pour leur permettre de protéger une position. je vous l'ai dit en débutant mon propos, cette situation devient malheureusement courante. J'ajoute que les fonctionnaires dotés de ce matériel sont formés et habilités. Ils doivent respecter un protocole précis, en termes de distance et de visée. Si ce protocole n'est pas respecté, c'est qu'un manquement est commis. Dès lors, il y a une enquête et le manquement doit être sanctionné. Puisque j'en viens à la question des fautes, j'aimerais dire deux choses.

En la matière, un certain nombre d'enquêtes ont été ouvertes ces dernières semaines auprès de l'Inspection générale de la police nationale et de l'Inspection générale de la gendarmerie nationale, notamment pour des faits allégués de mauvais usage de LBD. Au total, depuis le début du mouvement dit des « gilets jaunes », on compte environ 2 200 blessés parmi les manifestants et 83 enquêtes en cours à I'IGPN et à l'IGGN impliquant des faits qui ont fait intervenir des tirs de LBD. Chaque tir étant précisément enregistré, nous savons qu'il y a eu 13 095 tirs de LBD depuis le début du mouvement. Cependant, comme je vous le disais, cette Cependant, comme je vous le disais, cette arme n'est pas anodine et la sécurité de tous est notre priorité. C'est pourquoi nous avons pris des mesures. Ainsi, le ministre de l'intérieur a notamment exigé que tous les policiers et les gendarmes munis de LBD soient dotés de caméras-piétons pour pouvoir vérifier systématiquement le bon usage de l'arme et, surtout, contextualiser cet usage pour s'assurer qu'il a été effectué dans des conditions réglementaires. Certains posent néanmoins encore une question : pourquoi le choix du LBD ? D'abord, j'ai beaucoup entendu que le LBD était une forme d'exception française, une arme qui ne serait utilisée que dans notre pays : c'est faux ! D'autres polices l'utilisent. En Espagne, en Croatie, en Bulgarie ou encore en Slovénie, les forces de sécurité intérieures sont dotées de LBD.

à une situation particulière, dans des circonstances précises que les retours d'expériences ont permis d'identifier. Le LBD répond, dans ce cadre, à cet ancrage dans la violence de certains groupes d'émeutiers, à la multiplication des situations dans lesquelles les policiers ou les gendarmes se trouvent aux limites de de la légitime défense. Si nous supprimions les LBD, il ne resterait, dans bien des cas, que le corps à corps ou l'usage des armes de service. Je ne crois pas que nous souhaitions Mesdames, messieurs les sénateurs, j'aimerais que l'on ne se méprenne pas. S'il n'y avait pas de violences, il n'y aurait de blessés ni chez les manifestants ni chez les forces de l'ordre. Et pourquoi pas, pas de manifestation ! S'il n'y avait pas de casseurs, s'il n'y avait pas d'agresseurs, il n'y aurait aucun tir de LBD. S'il n'y avait pas de casseurs, s'il n'y avait pas d'agresseurs, il n'y aurait aucun tir de LBD. Très juste ! Je serai le premier à être rassuré lorsque les forces de l'ordre n'auront plus à utiliser les LBD. Cela voudra dire que les manifestations ont retrouvé leur calme et que les casseurs ont perdu.

Nous devons être vigilants et exigeants. Nous devons sans cesse vérifier que les règles d'emploi des LBD sont respectées, mais nous ne pouvons pas nous permettre de retirer à nos policiers et à nos gendarmes un moyen utile et nécessaire pour le maintien du bon ordre républicain.

Oui, cette doctrine a évolué depuis le 1 décembre, date à partir de laquelle nous avons été systématiquement confrontés à des individus violents qui commettent des exactions ! Les forces de l'ordre savent qu'elles ne doivent en tolérer aucune. Dès qu'il y a des violences, elles interviennent pour y mettre un terme. C'est ce qu'on attend d'une police et d'une gendarmerie républicaines, que vous appelez de vos voeux, madame Assassi.

la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui poursuit un objectif en partie légitime, celui de faire la lumière sur les conditions réelles d'utilisation des lanceurs de balles de défense dans le contexte des manifestations et les risques liés à cette pratique. Tel est l'objet de son article 2. Cet article fait directement écho aux objections que l'on a vu se multiplier ici et là, suite aux violences et aux dégradations qui ont été constatées lors des manifestations de « gilets jaunes Les préoccupations relayées par des institutions et des observateurs, comme le Défenseur des droits ou la Ligue des droits de l'homme, sont celles de nombreux de nos concitoyens désireux d'exercer leur droit de manifestation en toute sécurité. Elles doivent donc être entendues et prises en compte par les autorités chargées de maintenir l'ordre. Après un lent mouvement de pacification des cortèges, qui a participé à leur légitimation et leur a permis de peser dans l'histoire sociale de notre pays, nous observons, depuis quelques décennies, une recrudescence des violences liées aux manifestations, qui sont le fait de petits groupuscules violents. Il y a quelques années encore, le climat pacifique des mobilisations populaires était tel que l'on pouvait y apercevoir des familles, des enfants. Les bilans étaient plus au décompte des manifestants que des infractions constatées. Ce qu'on appelait hier les « ligues » sont devenues les « Black Blocs » aujourd'hui. Il s'agit d'individus bien entraînés, cagoulés et équipés d'objets susceptibles d'être utilisés comme des armes. Ils sévissent au milieu de manifestants pacifiques et provoquent nos forces républicaines. À ces comportements s'y agrègent d'autres plus erratiques, opportunistes, de casseurs et de pilleurs qui s'attaquent au bien public, au mobilier urbain et aux commerces. Pour qui n'a pas à endosser l'uniforme chaque samedi et à mettre en balance la protection de son intégrité physique, celle de ses collègues et l'utilisation d'armes engageant sa responsabilité personnelle et celle de l'institution policière, l'équation peut sembler simple. Nous tenons, au contraire, à réaffirmer notre confiance en nos forces de maintien de l'ordre et en leur sincérité à vouloir exercer leur mission dans l'intérêt de tous les Français, sans servir telle ou telle intention obscure. Il serait dangereux de laisser croire, comme le déclarait ironiquement Louis-Philippe, que « La République a de la chance, elle peut tirer sur le peuple ». Si la République n'a pas vocation à le faire, la désarmer pourrait la faire vaciller D'ailleurs, force est de constater que l'utilisation d'armes non létales est aujourd'hui plus polémique que celle d'armes létales. L'armement de forces de sécurités privées qui s'est renforcé sous le précédent quinquennat a suscité peu de réactions. Aujourd'hui, les alternatives ne sont malheureusement Du fait de cette contrainte, nous ne sommes pas favorables à une interdiction pure et simple des lanceurs de balles de défense, comme le dispose l'article 1 de la proposition de loi. Pour autant, le débat sur l'adaptation du maintien de l'ordre doit se poursuivre. Il devient urgent de retisser le lien entre les autorités et les services d'ordre des organisateurs de manifestations, lorsqu'ils existent, de même que les agents sur le terrain et les manifestants. La fragilisation des syndicats n'est pas un phénomène totalement étranger à la montée des violences que l'on observe dans les cortèges. Plusieurs de nos voisins européens ont expérimenté de nouvelles techniques ou outils de maintien de l'ordre visant à renforcer l'information des personnes manifestant pacifiquement, afin de permettre une interpellation plus efficace des individus violents. On pense, par exemple, au recours à des panneaux permettant de diffuser des messages de dispersion.

Les règles d'utilisation ont considérablement été renforcées par les instructions des 27 juillet et 2 août 2017 du ministre de l'intérieur, comme l'a noté le Conseil d'État dans son ordonnance du 1 février 2019. Depuis celle du 23 janvier 2019, s'y ajoute également l'obligation de filmer l'utilisation des LBD, obligation qui, sur le terrain, apparaît difficile à mettre en oeuvre. La création d'une commission d'enquête pour examiner ces questions aurait peut-être été plus pertinente. Le groupe du RDSE avait d'ailleurs déposé, en 2008, une proposition de résolution en ce sens s'agissant des Taser. C'est la raison

crains toutefois de vous déplaire en exposant l'avis que je formulerai tout à l'heure. Le texte proposé comprend deux volets principaux : la réflexion sur la mise en oeuvre de mesures alternatives à l'usage de la force dans les opérations de maintien de l'ordre et l'interdiction des lanceurs de balles de défense dans ce même cadre. Depuis quelque temps, dans le sillage des manifestations liées à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à la loi Travail et, plus récemment, du mouvement dit des « gilets jaunes », l'État est confronté à une augmentation significative des violences. Parfois très agressives, ces violences visant les biens, voire les symboles de la République, mais aussi les forces de l'ordre sont devenues récurrentes et, par moments, très provocatrices. Elles sont souvent le fait d'individus qui instrumentalisent dangereusement le droit à manifester et qui nuisent, par leurs actes, à l'image de ceux et celles qui expriment très légitimement, en manifestant, leurs revendications et opinions. Cette situation préoccupante conduit à s'interroger sur l'adéquation entre les pratiques actuelles du maintien de l'ordre pour prévenir les débordements et la nécessaire garantie du libre exercice du droit de manifester, eu égard à ce que je définirai comme la professionnalisation de l'affrontement violent et qui s'apparente à une forme de guérilla urbaine. Cette réflexion sur l'organisation des opérations doit naturellement intégrer une attention particulière aux conditions de l'octroi de l'habilitation

Je ne doute d'ailleurs pas, monsieur le secrétaire d'État, que face à la récurrence, à l'évolution de ces affrontements violents et de leurs formes, le Gouvernement n'ait déjà engagé une démarche d'évaluation. Le deuxième volet de cette proposition de loi porte sur l'interdiction de l'usage des lanceurs de balles de défense. Il convient de rappeler que les lanceurs de balles de défense constituent une arme de force intermédiaire à l'usage strictement encadré. Ils visent non le manifestant que je qualifierai « d'ordinaire », mais celui que j'appellerai le « fauteur de troubles ». L'usage de cette arme est conditionné à une absolue nécessité et à un déploiement proportionné. l'utilisation de ces armes, faut-il le rappeler, n'intervient que lors d'une situation extrêmement dégradée. Elle obéit à une procédure très spécifique. Il s'agit d'une arme de riposte et de défense qui ne peut être employée que pour disperser un attroupement, après des sommations prononcées par des autorités habilitées ou, à titre dérogatoire, lors de situations d'urgence ou d'agressions violentes qu'il n'est pas besoin ici de décrire, compte tenu des nombreuses images et scènes d'agressions violentes des agents des forces de l'ordre. Prévoir une interdiction de cette arme intermédiaire sans prévoir d'alternative est de nature à déstabiliser brutalement, soudainement et dangereusement l'organisation des opérations de maintien de l'ordre telles qu'elles existent aujourd'hui. En effet, retirer un échelon intermédiaire dans la palette des armes autorisées ferait forcément défaut dans la nécessaire gradation de la réponse que les forces de l'ordre se doivent d'apporter. On encourrait alors vraisemblablement deux écueils, qui sont le contraire de votre intention, madame la présidente Assassi : un risque de recours plus fréquent à une arme létale et une difficulté renforcée- et très sérieuse -à éviter le contact direct, souvent source de violences, entre forces de l'ordre et manifestants. Enfin, il apparaît que la plupart des dispositions proposées, en particulier l'article 1, relèvent non du domaine de la loi mais du domaine réglementaire. réglementaire. Il nous semble que cette proposition de loi n'est pas de nature à répondre à l'objectif annoncé : l'apaisement de l'organisation du maintien de l'ordre. Elle ne saurait davantage répondre aux formes d'agressions violentes très organisées auxquelles nos forces de l'ordre doivent faire face. Je citerai l'exemple des stages de formation à la guérilla urbaine, organisés à Notre-Dame-des-Landes par des zadistes, et qui posent question. Je voudrais redire ici le profond attachement des centristes au respect des libertés individuelles

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la situation sociale particulière dans laquelle se trouve notre pays ainsi que la multiplication des violences et des exactions en marge des manifestations des « gilets jaunes » ont occasionné depuis plusieurs mois un usage plus important des lanceurs de balles de défense dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre. La médiatisation de certains cas de blessures attribuées à l'utilisation de lanceurs de balles de défense, blessures que l'on ne peut que regretter, a conduit à une remise en cause de cette arme de force intermédiaire. Dès lors, s'interroger sur l'adéquation des dispositifs de maintien de l'ordre peut apparaître pertinent dans un contexte social et sécuritaire difficile. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi vise à interdire immédiatement l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre. Elle tend également à permettre une plus grande transparence des données relatives à l'usage des armes par les policiers : le lendemain de chaque manifestation durant laquelle les forces de l'ordre ont fait usage de leurs armes, le traitement relatif au suivi de l'usage des armes serait ainsi rendu accessible au public. Enfin, elle demande au Gouvernement la remise d'un rapport au Parlement qui serait « détaillé et documenté sur les avantages et les inconvénients de chaque type de doctrine type de doctrine au niveau européen, et sur les alternatives à mettre en oeuvre dans notre pays pour pacifier le maintien de l'ordre dans le cadre des manifestations ». Ce texte appelle toutefois un certain nombre de remarques. En premier lieu, lieu, il présente des difficultés d'ordre juridique. La plupart des dispositions de la proposition de loi ne relèvent pas du domaine de la loi. Les conditions d'emploi des armes dans le cadre des opérations de maintien et de et de rétablissement de l'ordre et la description des armes pouvant être employées sont définies par voie réglementaire. La liste des armes susceptibles d'être utilisées est ainsi fixée par décret. En deuxième lieu, l'article 2, qui ouvre au public le traitement relatif à l'usage des armes, présente un danger. En effet, non seulement cette disposition soulève des difficultés en termes de protection des données personnelles, mais elle pourrait également conduire à divulguer des données relatives aux conditions d'intervention des forces de l'ordre, risquant alors de fragiliser leur action. En dernier lieu, l'application de l'article 3, qui vise à repenser la doctrine française du maintien de l'ordre en s'inspirant des modèles mis en oeuvre par d'autres pays européens nécessite des travaux d'une certaine ampleur. Aussi, le délai de deux mois ne semble pas raisonnablement suffisant. En outre, notre doctrine française n'a rien à envier à celles qui sont mises en oeuvre au sein des autres pays européens. Pour preuve, nos agents de police et de gendarmerie nationales sont régulièrement sollicités par d'autres États de l'Union européenne afin de former leurs propres forces de maintien de l'ordre. Enfin, certaines pistes apparaissent plus pertinentes pour guider la révision de la doctrine française de maintien de l'ordre. Ainsi, renforcer la judiciarisation des actes de violence et de dégradation pourrait être privilégié. Monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la doctrine française de maintien de l'ordre repose sur un maintien à distance des individus commettant des exactions. Depuis plusieurs années, les lanceurs de balles de défense font partie intégrante de l'arsenal de maintien de l'ordre et leur usage est strictement encadré. Certes, l'utilisation de ces armes de force intermédiaire a récemment progressé dans de fortes proportions, mais cette augmentation s'explique par les violences sans précédent perpétrées à l'encontre des forces de sécurité intérieure dans le cadre des manifestations. Dès lors, pourquoi priver nos forces de l'ordre de l'usage d'une arme circonscrite à des finalités défensives et supprimer un échelon dans l'arsenal des moyens mis à leur disposition ? Pourquoi interdire l'usage de cette arme sans prévoir de la substituer par un autre équipement et prendre ainsi le double risque d'inciter au contact direct entre les manifestants et les forces de l'ordre et d'induire un recours plus fréquent à l'arme létale ? Pour toutes ces raisons, l'ensemble du groupe Les Indépendants ne votera pas en faveur de ce texte. La parole est à M. Alain Richard.

de contestation. Notre-Dame-des-Landes a été un marqueur très important du fait de sa durée et de la militarisation du comportement des occupants.

qui faisaient l'objet, j'y insiste, d'une régulation partagée. Car ces manifestations, qu'elles soient pilotées plutôt par des organisations, disons humanitaires ou de défense des droits de la personne, ou qu'elles soient proposées plutôt par des organisations syndicales, avaient

Ce à quoi nous devons maintenant nous confronter pour prendre des positions de responsabilités partagées en toute authenticité, c'est à la fréquence de manifestations qui débouchent sur des comportements

des « gilets jaunes » -, on observe un évitement de la faculté de déclaration de la manifestation et une défaillance quasi volontaire dans l'encadrement de ces manifestations. Il y a eu une

politiquement. Que faire ? Comment nous organiser ? Je me plais à constater qu'un grand nombre de représentants des différentes familles politiques du pays veulent participer et faire réussir le grand débat national, de manière à sortir de cette situation de confrontation de rue.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, permettez-moi de débuter cette intervention en vous citant quelques noms

front fracturé par un tir de LBD le 5 décembre ; Jérôme, quarante ans, éborgné par un tir de LBD le 26 janvier. On compte 1 700 blessés chez les manifestants depuis le 17 novembre, parmi lesquels 94 blessés N'oubliez pas les policiers ! Derrière l'impersonnel nombre des victimes, il y a des individualités, des vies, des quotidiens perturbés, des destins brisés par les violences policières. Ces LBD sont d'une extrême dangerosité : leur force d'impact est de 200 joules, soit l'équivalent d'un parpaing de vingt kilos qui vous serait lâché sur le visage à un mètre de hauteur. Ces armes mutilent, estropient et défigurent nombre de nos concitoyens, et souvent non pas parce que ceux-ci étaient responsables de violences, mais plutôt parce que le policier auteur du tir n'a le plus souvent pas employé son équipement de de manière adéquate. À l'échelon national, c'est la voix du Défenseur des droits qui s'est élevée pour alerter de la dangerosité des armes sublétales. À l'échelon supranational, c'est d'abord le Parlement européen qui a dénoncé la disproportion avec laquelle nos forces de l'ordre répriment les mouvements sociaux. Le Conseil de l'Europe a ensuite critiqué notre usage des LBD, contraire aux droits humains. Enfin, ce mercredi, c'est l'ONU, par la voix de sa haut-commissaire aux droits de l'homme, qui demande une enquête approfondie sur les cas d'usage excessif de la force sur le sol français. Alors qu'il devait à l'origine être employé dans des contextes de guérilla urbaine, le lanceur de balles de défense est aujourd'hui abusivement utilisé lors de manifestations. En partant de ces constats, nous proposons l'interdiction immédiate du recours aux LBD dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre, ainsi

Nos voisins ne font-ils pas face à des violences citoyennes, notamment en Allemagne avec l'infiltration de néonazis dans les cortèges ? Pourtant, nombre de nos partenaires européens ont choisi une approche différente dans la gestion des violences. Ainsi, en Allemagne, enseigne-t-on aux forces de l'ordre la philosophie de la « désescalade Celles-ci agissent en amont, afin de prévenir toute atteinte à l'ordre public. Chez nous, on laisse les Black Blocs et autres minorités violentes proliférer dans les cortèges avant d'intervenir une fois les méfaits commis. S'ensuivent alors des répressions généralisées sans la moindre distinction entre manifestants et casseurs. En termes d'arsenal, alors que nous utilisons des armes susceptibles de blesser nos concitoyens, les Allemands se limitent à des dispositifs permettant de garder les foules à distance. De surcroît, nos méthodes pour contenir les violences créent une promiscuité oppressante, dont le nassage, qui ne peut qu'engendrer une escalade de la brutalité entre policiers ces derniers étant encerclés de toutes parts et n'ayant même pas la possibilité de quitter la manifestation par une rue adjacente.

en Hollande ou des « officiers de dialogue » en Suède. Il est d'ailleurs à noter que ces deux pays possèdent des forces de police presque désarmées et sont pourtant considérés comme plus « sûrs » que la France par le World Economic Forum. Preuve s'il en est que ce n'est pas par l'armement dissuasif qu'on instaure la paix sociale. Prenant acte de ces différences, nous demandons au Gouvernement la remise d'un rapport sur les différentes doctrines

Une meilleure formation des gardiens de la paix et un meilleur encadrement de leurs pratiques seraient un premier pas pour éviter que, à l'avenir, de nouvelles violences incontrôlées ne soient perpétrées. Tirons des leçons des événements tragiques du passé, dont les morts de Malik Oussekine et de Rémi Fraisse. Cette proposition de loi n'est pas une offense faite aux forces de l'ordre

la nécessité du maintien de l'ordre public et, dans le même temps, la nécessaire garantie des libertés publiques, notre groupe défendra trois idées fortes. Nous exprimons d'abord un soutien sans réserve aux forces de l'ordre, engagées depuis plusieurs années, sur tous les fronts, dans des opérations complexes et usantes de maintien de l'ordre face au terrorisme, face à un regain des formes radicales de violence dans les manifestations. Nous voulons aussi affirmer que la gravité des lésions suscitées par l'usage des LBD a atteint un niveau insoutenable pour notre société. Enfin, nous adhérons à l'idée défendue par nos collègues communistes l'usage des LBD doit être prohibé dans le cadre du maintien de l'ordre et que des alternatives à cette arme doivent être recherchées au plus vite. Le texte qui nous est proposé permet d'aborder une partie des problématiques de sécurité dans le pays en ce qui concerne le maintien de l'ordre. Il est difficile de décorréler son examen de la proposition de loi Retailleau-Castaner dont nous débattrons mardi. S'agissant du texte de Mme Assassi, je tiens à saluer la position défendue par Mme la rapporteure, qui n'est pas dans le déni. En effet, celle-ci relève les possibilités d'amélioration en matière de formation des forces de l'ordre. Les Les syndicats des forces de l'ordre que nous avons auditionnés ont également insisté sur ce sujet, à tel point que nous nous interrogeons sur le rôle que les sénateurs pourraient jouer sur cette question. La rapporteure a raison quand elle pointe certains éléments d'imprécision juridique de la proposition de loi de Mme Assassi. Ce texte relève-t-il du domaine réglementaire ou du domaine législatif ? Je considère, pour ma part, qu'il relève avant tout du politique ! Premier constat, chers collègues : la confiance de nos concitoyens envers la police reste largement majoritaire. La marche pour la paix du 11 janvier 2015 avait parfaitement symbolisé cette relation avec des images remarquées d'hommage aux forces de l'ordre. Le Cevipof nous indique que la confiance de la population française envers la police est en légère hausse et s'élève à 74 % en 2018. Plusieurs facteurs objectifs ont sans doute participé au réchauffement des relations entre la police et la société lors du dernier quinquennat le nouveau code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie, entré en vigueur en 2014, a ainsi rendu obligatoire le port du matricule et encadré les palpations de sécurité. Rappelons d'ailleurs que c'est un autre socialiste qui avait mis en place le premier code de déontologie, le toujours respecté Pierre Joxe. En juin 2016, toujours sous François Hollande, une expérimentation autour du port de mini-caméras a été lancée au sein de la police municipale. L'augmentation des effectifs, après un quinquennat Sarkozy qui les avait vus fondre de 12 000 hommes et femmes, a également constitué un complément nécessaire à ces mesures d'apaisement. Durant la campagne de 2017, Emmanuel Macron avait donné l'impression de vouloir poursuivre sur cette voie, combinant à la fois le renforcement des moyens dédiés à l'amélioration des conditions de travail de nos forces de police et de gendarmerie et, « en même temps », l'amélioration des relations entre policiers, gendarmes et citoyens. Ainsi, promesse a été faite de recruter 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires ; ces moyens supplémentaires ont été accompagnés d'une nouvelle police, dite « police de sécurité du quotidien », supposée être de proximité, mais à la création de laquelle la population n'a guère été associée. Ces promesses relevaient de bonnes intentions, mais, comme souvent dans le monde macroniste, la traduction en actes et l'accompagnement politique ont failli. Ainsi, les nouveaux moyens humains alloués ne satisfont que partiellement les besoins des forces de l'ordre. Comme l'a très richement documenté la commission d'enquête sénatoriale relative à l'état des forces de sécurité intérieure, les mesures ponctuelles prises ces dernières années n'ont pas enrayé la dégradation continue des conditions matérielles de travail- équipement et immobilier -des forces de sécurité intérieure ». Il faut rappeler ici les conditions d'exercice des missions de maintien de l'ordre. Que nous disent les policiers ? Des stands de tir parfois hors d'âge, des conditions d'entraînement dégradées, même dans la région parisienne, des heures de formation insuffisantes et pourtant difficiles à consommer, ou encore la nécessité, notamment en province, de faire les « fonds de tiroir » en termes d'effectifs et de moyens matériels, quitte à mobiliser dans les manifestations des agents insuffisamment formés et sous-équipés. Des fonctionnaires de police nous racontaient hier encore comment un gradé avait dû aller chez Decathlon acheter sur ses fonds propres des casques et des genouillères pour ses hommes, faute d'équipements adéquats. Aussi, l'objectif d'amélioration du lien police-population, passé au second plan dans le débat public dans le contexte terroriste, nous semble aujourd'hui nécessiter un traitement prioritaire. Les forces de l'ordre ont le sentiment d'être trop souvent pointées du doigt en cas de bavure supposée et trop peu soutenues en cas de violences dirigées contre elles. Avec le groupe socialiste, nous avons rencontré hier des syndicats de forces de l'ordre. Ils nous ont indiqué que la première personne à avoir perdu l'usage d'un oeil dans le mouvement dit des « gilets jaunes » était un policier. que membres d'un parti de gouvernement, nous sommes pleinement conscients des exigences auxquelles ils sont soumis quotidiennement, de la mobilisation usante qu'ils assurent chaque week-end, du sacrifice qu'ils font pour protéger directement la République, ses symboles et ses représentants. Parallèlement, et c'est évidemment le coeur de cette proposition de loi, nous avons une claire conscience des violences subies par certains de nos concitoyens civils. Documentées pour beaucoup sur les réseaux sociaux pendant la mobilisation des « gilets jaunes », celles-ci sont restées absentes du champ médiatique pendant plusieurs semaines. L'accumulation malheureuse de ces violences a conduit journaux et télévisions à aborder le sujet en ce début d'année 2019. Le ministre de l'intérieur, qui indiquait jusqu'à il y a peu qu'il ne connaissait aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des « gilets jaunes », a finalement consenti à équiper de caméras les policiers chargés de tirer avec des lanceurs de balle de défense. Cette première avancée est-elle suffisante ? On peut en douter, puisque des blessures graves provoquées par des LBD ont continué d'être recensées. Le déni permanent de l'existence de difficultés de relations entre la police et la population est dangereux. Il laisse s'installer dans la population un ressentiment qui se retourne contre les forces de l'ordre, alors même que ces dernières ne disposent pas de toutes les cartes en main pour changer la situation. La solution doit aussi, si ce n'est surtout, venir de la discussion politique. À ce titre, nous regrettons que cette question des relations entre les forces de l'ordre et la population soit absente du grand débat national, alors même qu'une partie de la population a été confrontée à la problématique du maintien de l'ordre pour la première fois à l'occasion du mouvement des « gilets jaunes Au-delà de cet épisode des « gilets jaunes », qui ne couvre pas tout le spectre des relations entre la police et la population, notre pays mérite un débat serein sur la confiance que la police lui inspire et les moyens de l'améliorer. Les Français ont le droit d'être exigeants avec leur police. Ils ont le droit de s'interroger sur l'opportunité d'engager des unités peu habituées au maintien de l'ordre sur le terrain. Avec mes collègues socialistes, nous avons hésité sur la position à adopter quant à cette initiative. Les prises de position successives et contradictoires d'anciens ministres, d'experts, de chercheurs sur le maintien de l'ordre, de journalistes, d'ONG, de policiers ou d'institutions internationales appellent à l'humilité : le sujet est complexe, nous le savons. L'exercice du maintien de l'ordre est un art délicat. L'exercice des fonctions de ministre de l'intérieur n'est pas davantage une sinécure dans un contexte social français actuel, qui n'est pas indifférent. Des blessés dans les manifestations, il y en a dans tous les pays. Des blessures irréversibles, c'est plus rare ! Et c'est bien ce qui pose question avec les LBD Le docteur Laurent Thines, professeur de neurochirurgie au CHU de Besançon, a ainsi lancé une pétition pour un moratoire sur l'utilisation des armes sublétales, afin d'alerter « sur leur dangerosité extrême ». Rien ne justifierait de telles blessures irréversibles face à des casseurs ; rien ne justifierait de telles blessures face à de simples manifestants innocents. C'est sans doute ces blessures graves qui ont attiré l'attention d'organisations internationales. Les demandes du Défenseur des droits, du Conseil de l'Europe et des Nations unies ne peuvent être balayées d'un simple revers de la main. On ne peut pas appeler à une renaissance de l'Europe, tout en se moquant d'une résolution du Parlement européen. Face au déni qui semble caractériser l'exécutif sur ces questions de libertés publiques, nous avons décidé de tirer la sonnette d'alarme. C'est pourquoi nous voterons le texte de nos collègues communistes, quand bien même il présente des imperfections. C'est pour nous un moyen d'appeler au débat sur la formation des forces de l'ordre, leur doctrine d'emploi, l'accent à mettre sur la recherche d'alternatives aux LBD. Après les manifestations contre la loi El Khomri, une commission d'enquête à l'Assemblée nationale avait également évoqué cette piste indispensable, cherchant par exemple des solutions du côté de systèmes lumineux produisant un éblouissement non vulnérant, ou de systèmes sonores diffusant des messages ou utilisant des fréquences provoquant un inconfort. Derrière l'usage des LBD, et leur incontestable et insupportable dangerosité, nous ne pourrons pas éviter plus longtemps le débat crucial sur les moyens et la doctrine d'emploi de nos forces de l'ordre. Oui, les policiers doivent avoir les moyens de se protéger Oui, il faut condamner les violences des extrémistes et des casseurs ! Mais non, cela ne peut suffire à accepter des dommages collatéraux ! Les journalistes et manifestants pacifiques qui ont essuyé des tirs de LBD ne le comprendraient pas. Surtout, cela nuirait à terme à la fois à la bonne image et au respect qui sont dus à nos forces de police. La parole est à M. François Grosdidier.

C'est vraiment la dernière chose à faire au moment où les forces de l'ordre n'ont jamais été autant agressées, aussi violemment, et le plus souvent gratuitement. Nous avions pu le constater, unanimement d'ailleurs, madame Assassi, lors des travaux de la commission d'enquête sur l'état des forces de sécurité intérieure. Non, le problème de la France de 2019 n'est pas la violence policière, même si MM. Poutine et Erdogan s'en inquiètent ! C'est l'ONU qui s'en inquiète ! Non, le problème de la France de 2019, c'est bien la violence contre les policiers

c'est même plutôt le contraire ! Le problème de la France de 2019, c'est bien la violence de plus en plus débridée, une violence qui atteint même les agents des forces de l'ordre. Ceux-ci, par discipline et par éthique, s'imposent une réponse proportionnée.

la réponse aura d'ailleurs été plus insuffisante qu'excessive, puisque l'État n'a pas pu complètement la juguler et, en tout cas, pas rapidement. La doctrine française du maintien de l'ordre visait d'abord à contenir les manifestations et à éviter le contact. Mais cela valait

? Le LBD est indispensable, non comme outil de maintien de l'ordre, mais comme réponse aux délinquants, qui doivent être neutralisés de la façon la moins dommageable pour eux-mêmes. Bien sûr, et sur ce point

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la France vit une période intense- c'est peu de le dire -en matière d'ordre public. Nos gendarmes et nos policiers sont particulièrement mobilisés à ce titre : interventions dans les ZAD pour rétablir l'ordre, mouvements socioprofessionnels et, enfin, crise des « gilets jaunes » exceptionnelle par son ampleur, comme par sa durée. Le recours accru à la violence par une frange radicale d'opposants apparaît de plus en plus systématique. La présence de groupes d'individus, venus à la seule fin d'en découdre avec les forces de sécurité intérieure, est un phénomène de plus en plus récurrent. Provenant pour la plupart de mouvements ultras, ces individus intègrent les manifestations, afin d'y provoquer des incidents avec les forces de sécurité intérieure. Équipés de casques, de masques respiratoires et de protection, souvent armés et parfaitement organisés, ces individus cherchent l'affrontement. Ainsi, 1 430 policiers et gendarmes ont été blessés depuis le 17 novembre. Et combien de commerces pillés, combien de voitures et de biens privés saccagés ? Mêlés à la foule des manifestants, ces voyous créent un climat délétère et cherchent à entraîner dans les affrontements d'autres catégories de personnes. Nos forces de sécurité sont donc aujourd'hui confrontées à un défi paradoxal assurer le bon déroulement de manifestations, afin de protéger les participants et les tiers, d'une part, et répondre de manière proportionnée et ciblée au déchaînement de violence, d'autre part. Notre dispositif actuel de maintien de l'ordre est efficace pour répondre à ces enjeux parfois contradictoires. Il pourrait se résumer en quatre points clés : primat de l'autorité civile, seule habilitée à décider de l'emploi de la force gradation dans l'emploi de la force avec une palette de moyens permettant de répondre à tous les scénarios, du service d'ordre paisible jusqu'au rétablissement de l'ordre insurrectionnel maintien à distance des opposants, afin d'éviter les affrontements au corps à corps, dangereux pour les forces de sécurité, comme pour les opposants ; déploiement d'unités spécialement formées et entraînées au maintien de l'ordre. La proposition de loi que nous examinons a pour principal objet d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense. Il s'agit d'une idée démagogique et dangereuse. Le LBD 40 est un outil utile pour maintenir à distance des adversaires dangereux et agressifs qui, parce qu'ils portent des masques, sont particulièrement immunisés contre les gaz lacrymogènes et qui veulent s'approcher, soit pour lancer des projectiles sur les forces de l'ordre, soit pour les agresser avec des armes blanches. Le LBD 40 n'est pas prévu pour disperser un attroupement. Il n'est utilisé que pour se défendre face à des individus violents qui agressent les militaires ou cherchent à s'emparer d'un point ou d'un monument que ceux-ci ont à défendre. Son emploi est strictement encadré.

qui n'a reçu qu'un signalement relatif à l'usage d'un LBD sur un total de trente-six signalements reçus depuis le début de la crise. À ce jour, le LBD est un outil indispensable à la réussite de manoeuvres d'ordre public sensibles, qui est éprouvé depuis plus de dix ans. En priver les forces de sécurité conduirait à les désarmer partiellement face à des individus violents, face auxquels le contact physique rapproché deviendrait l'unique solution. Par ailleurs, les forces de sécurité intérieure ne pourraient plus dissuader les individus porteurs de projectiles particulièrement dangereux de les approcher. Personne ne souhaite que nous en arrivions là. Les conclusions récentes du Conseil d'État, saisi au sujet de l'emploi du LBD dans le cadre du maintien de l'ordre, vont d'ailleurs dans ce sens. J'ajoute que chaque blessure fait évidemment l'objet d'une enquête interne, assortie d'une sanction lorsqu'une faute est

À ce sujet, je note que l'on envoie trop souvent, pour sécuriser des manifestations où figurent des individus potentiellement violents, des agents insuffisamment formés, par contraste avec les gendarmes mobiles ou les CRS. Cela tient essentiellement à une cause : à force de vouloir jouer la sécurité sociale du monde entier, l'État n'exerce plus correctement ses missions régaliennes ! Par ailleurs, il faut bien le dire, il existe une curieuse complaisance envers les casseurs d'extrême gauche. Comment peut-on expliquer, sans cela, que des individus notoirement violents et parfaitement identifiés puissent, sans la moindre difficulté, se joindre aux cortèges pour casser et piller ?

avec des blessures plus graves et plus nombreuses. De même qu'il est absurde de suspendre les libertés de tous les citoyens, au motif que certains d'entre eux sont violents, il est absurde d'empêcher les forces de l'ordre de se défendre parce que les LBD sont parfois, très rarement, utilisés à mauvais escient.

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, symboles de la République vandalisés, vitres de l'hôpital Necker brisées, scènes de guérillas urbaines inédites ... Qui n'a pas été choqué par ces actes insensés qui se déroulent dans nos rues ?

Dorénavant, chaque semaine, nos forces de l'ordre font face, avec courage et détermination, en tentant d'éviter le pire, qui peut arriver à tout moment. Je tiens à leur rendre hommage, manière que j'ai une pensée pour tous les blessés des manifestations, indépendamment de leur camp. Dans ce contexte, il est donc proposé, ici, d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense, autrement dit de priver les forces de l'ordre d'une arme, sans leur proposer aucune solution alternative.

Ses conditions d'utilisation sont d'ailleurs très strictes : en cas de légitime défense, face à un danger imminent ou si des violences sont exercées à l'encontre des forces de l'ordre. Ensuite, le lanceur de balles de défense est une arme intermédiaire, après l'emploi des armes non létales et avant qu'une arme létale puisse être utilisée après sommation. La Cour européenne des droits de l'homme exige que chaque pays soit équipé d'un arsenal gradué. Supprimer le LBD renforcerait donc le risque d'usage disproportionné de la force publique et augmenterait très sensiblement le nombre de blessés, d'autant que le maintien de l'ordre passerait d'une doctrine du maintien à distance au profit du corps à corps.

nécessaire au maintien de l'ordre public compte tenu des circonstances, et, d'autre part, proportionnée au trouble à faire cesser ». Non, cette arme n'est pas une atteinte au droit de manifester ! Elle s'adresse, en premier lieu, à ceux qui veulent en découdre avec la police ou la gendarmerie, aux casseurs qui n'ont aujourd'hui plus de limites. Qu'en est-il du droit des forces de l'ordre de se défendre en dernier recours, mais aussi de protéger la liberté des personnes désireuses de manifester pacifiquement ? Non, cette arme n'est pas disproportionnée ! Je ne crois pas que nos policiers tirent pour le plaisir. Les situations d'extrême tension, où les cibles sont mouvantes et au cours desquelles ils peuvent craindre pour leur vie, commandent de repousser les assaillants ultraviolents. Non, je n'ignore ni les blessures d'une particulière gravité de certains manifestants ni les erreurs qui ont pu être commises, pouvant donner lieu à des enquêtes approfondies et des sanctions exemplaires d'une très grande fermeté, d'ailleurs sans que l'on ait attendu les injonctions inadmissibles de l'ONU ! Dans ce cadre, je suis tout à fait favorable au renforcement de la formation des policiers et des gendarmes à l'usage de cette arme. Celle-ci contribue à faire respecter l'ordre républicain. Or, sans ordre républicain, le contrat social est rompu et la République est en danger. l'usage des LBD participe donc au renoncement de l'autorité de l'État, et je ne peux m'y résoudre. Pour toutes ces raisons, je voterai contre cette proposition de loi.

Jean-Pierre Grand. L'article 1 de la proposition de loi a pour objet d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense, appelés communément flash-ball, dans le cadre du maintien de l'ordre. Depuis des semaines, nos forces de l'ordre sont mobilisées et durement éprouvées.

De nombreuses vidéos en ligne en témoignent, sans pour autant montrer objectivement les longues minutes qui précèdent, pendant lesquelles nos forces de l'ordre font preuve d'un sang-froid exemplaire, malgré les provocations et les affrontements avec des individus déterminés à blesser, voire à tuer leurs membres. Dans ses Dans ses décisions récentes, le Conseil d'État a considéré que ces armes demeurent particulièrement appropriées pour ce type de situations. Je vous propose donc, mes chers collègues, de supprimer l'article J'aurai l'occasion, si nous allons plus loin dans la discussion, de revenir dans quelques instants sur la problématique des sommations, sous-jacente à cette initiative parlementaire. Quel est l'avis de la commission ? Dans la mesure où la commission des lois s'est prononcée contre la proposition de loi, l'avis est favorable

Le scrutin est ouvert.

si celui-ci n'était pas adopté, il n'y aurait plus lieu de voter sur l'ensemble de la proposition de loi, dans la mesure où les trois articles qui la composent auraient été supprimés. Il n'y aurait donc pas d'explication de vote sur l'ensemble. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Nous voterons donc contre la suppression de cet article et nous aurions voté pour la proposition